Madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, lundi, aux premières heures du jour, jour, un tremblement de terre a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. Il a été suivi de nombreuses et violentes répliques. Alors que le bilan humain de cette catastrophe s'alourdit de jour en jour, nos premières pensées vont aux victimes et à leurs proches, ainsi qu'aux équipes mobilisées pour leur porter secours. Nous serons attentifs à ce que tous les secours nécessaires parviennent aux populations touchées, où qu'elles se trouvent et sans autre critère que celui de l'urgence. Nous serons

Mme la Première ministre. Dès lundi, le Président de la République a annoncé la mobilisation de notre pays et proposé une aide d'urgence. Des sapeurs-pompiers, des sapeurs-sauveteurs et des personnels du centre de crise et de soutien sont arrivés sur place. Ils contribuent aux recherches sur le terrain. Pour aider les blessés, nous avons également proposé l'envoi d'un hôpital de campagne de la sécurité civile.

Depuis la privatisation, c'est le même constat : profits démesurés, péages toujours plus chers ! En revanche, ce qui est nouveau, c'est que désormais, au sein même de Bercy, ce constat interroge et même, d'une certaine façon, scandalise. La presse s'est ainsi fait l'écho d'un rapport de 2021 très instructif de l'inspection générale des finances. Il explique que ces entreprises ont une rentabilité très supérieure à celle qui

Les sommes en cause permettraient une réduction de près de 60 % des péages ou un prélèvement allant jusqu'à 55,4 milliards d'euros pour l'État- une paille

comment justifiez-vous que l'État ne fasse pas tout pour faire baisser les péages et mettre fin aux concessions actuelles ? Êtes-vous prêt à travailler avec le Parlement sur l'hypothèse d'une renationalisation ?

de la décarbonation des transports- reports fluviaux, investissements dans le ferroviaire, etc. Dépenser de l'argent pour racheter les autoroutes irait à l'encontre de la transition écologique et se traduirait à la fin par une mauvaise allocation des ressources publiques.

en faveur des industries et de la décarbonation, mais avec un double risque : des subventions massives attribuées de façon discriminatoire contre les vendeurs européens et une attraction potentielle

Quel bilan tirez-vous de vos discussions avec les autorités de Washington ? Quel aboutissement pensez-vous obtenir très prochainement en faveur d'un réarmement industriel européen ? de traiter de façon dynamique deux sujets bien connus entre Européens : les règles de concurrence interne et les aides d'État. Il reste un sérieux effort de convergence entre Européens à fournir d'ici au sommet prévu demain et après-demain, si nous

La première conclusion, cela ne vous surprendra pas, c'est l'efficacité du couple franco-allemand et l'alignement entre l'Allemagne et la France sur la nécessité d'accélérer nos investissements en matière de décarbonation industrielle et d'industrie verte. De ce point de vue,

nos alliés américains sont prêts à des ouvertures. Ils en ont d'ailleurs fait pendant notre déplacement. Ainsi, ils sont prêts à des ouvertures pour inclure un certain nombre de biens industriels européens : les voitures électriques dans le cadre du et des véhicules commerciaux,

sur le montant des subventions et des aides, ce qui est indispensable pour garantir une concurrence équitable, et ils sont prêts à ce que nous préservions nos investissements stratégiques. La troisième conclusion, la plus importante,

doit nous permettre de rivaliser à armes égales avec les États-Unis. Je souhaite que, au prochain Conseil européen- c'est la position que défendra le Président de la République -, nous puissions mettre en oeuvre sans délai le projet de la Commission européenne de façon à ce que nous soyons capables d'accélérer la réindustrialisation de l'Europe et la décarbonation de notre industrie. Il y va de notre souveraineté et de notre indépendance. Il existe encore- -des divergences de vues entre Européens. Il faut les surmonter : c'est la condition pour que l'Europe continue de jouer les premiers rôles en matière industrielle au XXI siècle. La parole est à M.

Madame la Première ministre, elle s'appelle Véronique, elle a 53 ans, je l'ai rencontrée hier lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Après deux années d'apprentissage en charcuterie, Véronique a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Pendant de longues années, elle a trimé sur les marchés, dans le froid de l'hiver, parfois jusqu'à-12 degrés, en soulevant de lourdes charges, si bien qu'à seulement 33 ans elle a dû se faire opérer de la colonne vertébrale. Malgré cette vie de labeur, malgré la pénibilité de son travail, avec les arrêts maladie et les périodes de chômage, Véronique ne pourra partir à la retraite qu'après avoir cotisé 44 années ! C'est plus que vous et moi, qui ne subissons pas la pénibilité physique de son travail.

c'est à toutes les Véronique de France que vous en faites payer la facture ! Aujourd'hui même, on apprend que l'entreprise Total a réalisé en 2022 des profits record : 19,1 milliards d'euros ! C'est plus que les 13,5 milliards d'euros de déficit que vous prévoyez pour le système de retraites à l'horizon de 2030. Alors, madame la Première ministre, quand allez-vous taxer ces superprofits ? Quand allez-vous écouter les centaines de milliers de Françaises et de Français qui étaient hier dans la rue pour dire non à la retraite à 64 ans ? Quand allez-vous retirer ce projet injuste et brutal ?

par rapport à la situation actuelle il n'est pas impossible que sa situation personnelle s'en trouve améliorée ! Eh oui ! Alors, tout va bien ! Monsieur le sénateur, vous parlez de Véronique comme étant exposée à des températures extrêmes.

amené à voter lorsque j'étais député socialiste. À l'époque, la gauche de gouvernement ne reniait pas les fondamentaux qui étaient les siens, à savoir être capable de prendre des décisions, même difficiles, quand il fallait conforter notre modèle social, et être capable de prendre des décisions favorables à l'emploi. Cette gauche que j'ai connue et que j'ai quittée- je dois vous dire que je n'en ai pas de regret aujourd'hui Nous non plus ! ... était capable de s'enthousiasmer, lorsque des entreprises créaient de la richesse et de l'emploi dans le pays. Nous célébrions l'idée qu'un jour nous puissions inverser la courbe du chômage. Il est vrai, monsieur le sénateur, qu'il a fallu attendre 2017 pour que cette fameuse courbe s'inverse. Cela vous peine peut-être à titre personnel, mais, comme vous servez, j'en suis sûr, l'intérêt général, l'intérêt général, vous devriez avec notre majorité vous en réjouir ! Enfin, monsieur le sénateur, ne me dites pas que vous confondez sciemment le bénéfice mondial d'un groupe international avec le financement

Monsieur le ministre, nous n'avons pas de leçon à recevoir d'une personne qui a avoué avoir voté pour Nicolas Sarkozy en 2007 ! Qui plus est, je tiens à rappeler

ayez le courage de revenir sur les exonérations de cotisations patronales qui sont inefficaces et coûteuses, de contraindre les entreprises à améliorer leur taux d'emploi des seniors et surtout de taxer les superprofits- taxez-les et on pourra financer les retraites

Après l'adoption définitive, hier, du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, je souhaite alerter, une nouvelle fois, le Gouvernement sur les dysfonctionnements de certains dispositifs de transition écologique. Une nouvelle fois, car je l'avais déjà interpellé sur ce sujet en novembre dernier. Certes, chaque collectivité, entreprise, citoyen, est acteur du changement climatique, mais l'État, par sa puissance d'impulsion et d'action, a un rôle primordial à jouer. Aussi, il est d'autant plus dommageable de constater que des dysfonctionnements majeurs subsistent, notamment dans l'application du dispositif MaPrimeRénov'. Je ne compte plus les alertes reçues à ce sujet- et je sais qu'il en est de même pour bon nombre de mes collègues -de la part de particuliers, d'artisans, mais aussi de maires qui font remonter les inquiétudes de leurs administrés. Trois éléments principaux sont en cause. D'abord, la complexité du dispositif et du site internet, y compris pour des personnes qui sont à l'aise avec l'outil informatique. peuvent se passer pour les 14 millions de Français qui souffrent d'illectronisme ! Ensuite, les délais, qui peuvent atteindre plusieurs mois, pour recevoir une subvention parfois très en deçà de ce qui avait été annoncé. avons tous été sensibilisés par des particuliers qui avaient reçu des sommes bien inférieures à celles qui leur avaient été promises, et ont ainsi été dans l'obligation d'emprunter pour compenser la différence. Enfin, les entreprises attendent parfois le versement de la prime pour faire payer le client, ce qui les met, elles aussi, dans une situation délicate. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) indique même que certaines entreprises se trouvent confrontées à des négociations difficiles avec les banques et qu'elles sont sans ces entreprises, l'ambition du Gouvernement en matière de transition énergétique est vaine. Aussi, j'aimerais connaître les actions engagées pour améliorer le dispositif et le rendre, enfin, pleinement opérationnel.

lors de ses voeux, en 2021, le Président de la République louait les première, deuxième et troisième lignes qui avaient tenu notre pays durant la pandémie. Parmi ces engagés, ces solidaires, se cachent votre soeur, votre voisin, vos amis, des milliers d'anonymes, nous disait-il. Marie, infirmière, Fouad, animateur, Rosalie, vendeuse, Thibaud, agent d'entretien, Florence, auxiliaire de vie, etc. : ces héros de notre République étaient hier dans la rue, ils y seront samedi et les jours suivants, ils ne lâcheront pas ! Ils ne lâcheront pas, car ils ne comprennent pas votre acharnement à leur prendre deux années de leur vie. Ils ne lâcheront pas, car ils ne comprennent pas vos contradictions. Ils ne lâcheront pas, car ils ne comprennent pas le sens de votre obstination. Et je l'avoue, madame la Première ministre, je ne vous comprends pas non plus : rien de tout cela ne vous ressemble. Vous nous disiez lors de votre déclaration de politique générale : « Les Français ont élu une Assemblée sans majorité absolue. Ils nous invitent à des pratiques nouvelles, à un dialogue soutenu et à la recherche active de compromis. Les pratiques nouvelles ? Le 47-1 ! Le dialogue ? Le 49.3 ! Les compromis ? « C'est non négociable » ! En résumé : déni, mépris ! Madame la Première ministre, vous savez que l'on ne gouverne pas contre le peuple. Cessez d'appliquer une consigne que vous savez absurde, cessez de vouloir passer en force, cessez d'ignorer les syndicats, les parlementaires et le peuple, cessez d'ignorer une société qui change ! Marie, Fouad, Rosalie, sont fatigués, mais ils ne lâcheront pas. Ils ne lâcheront pas, parce que leur combat est juste- et vous le savez. Une seule question les taraude : quand ? Quand allez-vous retirer ce projet de loi aussi inutile qu'injuste ?

une fois de plus, vous avez multiplié les phrases définitives et les caricatures ... Alors, une fois de plus, dans un esprit de responsabilité, je veux vous rappeler les faits

La question qui se pose au sujet de cette réforme est la suivante : voulons-nous, oui ou non, conserver notre système de retraite par répartition ? Pour y parvenir, il est vrai que nous demandons un effort aux Français. C'est le seul chemin pour assurer l'équilibre de nos retraites. Ce chemin, le Sénat ne le découvre pas.

monsieur le président Gontard, je mesure parfaitement ce que travailler plus longtemps représente pour beaucoup de Français. C'est pourquoi nous avons mené, pendant plusieurs semaines, des concertations avec les organisations syndicales et patronales, ainsi qu'avec les groupes parlementaires. : aux termes de notre projet, quatre Français sur dix- ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui exercent des métiers pénibles -n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans. Alors, je ne doute que Fouad, Marie et Rosalie font partie de ces Français qui n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans. Or que proposez-vous à ces Français, monsieur Gontard ?

de cible, car les plus riches auront toujours une retraite, même sans notre réforme. En revanche, pour les classes moyennes, pour les plus modestes, ce serait plus de chômage et moins de pouvoir d'achat. Ce que nous proposons, c'est le plein emploi et de meilleures retraites

Il évoluera et s'enrichira encore grâce au débat parlementaire. Certes, je sais que la dirigeante de votre parti a appelé à faire du Parlement une « zone à défendre », une ZAD, mais j'ai confiance dans la responsabilité de chacun pour offrir aux Français un débat de bonne tenue, un débat d'idées, un débat respectueux. Je ne doute pas que le Sénat y sera particulièrement attentif. La parole

Territoires. Monsieur le ministre, l'éducation nationale vient d'informer de nombreux maires ruraux de projets de fermeture de classes, sans qu'ils aient été préalablement consultés. À titre d'exemple, en Loire-Atlantique, 29 communes rurales ont une épée de Damoclès au-dessus du toit de leur école. école. Les écoles rurales sont le théâtre d'un drame qui se joue année après année. Les fermetures de classes pénalisent les familles, obligées de réaliser de plus longs trajets. Elles privent les petites communes d'un élément central de leur vitalité et de leur attractivité. Le Président de la République avait assuré, en 2019, qu'aucune classe ne fermerait sans l'accord du maire de la commune. Récemment, votre ministère s'est engagé à mieux prendre en compte les contraintes territoriales. La méthode actuelle de gestion de la carte scolaire n'est pas adaptée aux réalités du monde rural. Les décisions d'ouverture ou de fermeture de classes ne sont-elles pas prises, chaque année, un peu trop tôt pour la rentrée suivante Il est regrettable de ne pas se projeter à moyen terme, alors que de petites communes consentent de lourds investissements financiers pour mettre aux normes des locaux scolaires. Les élus naviguent à vue et ont le sentiment que le nombre de professeurs disponibles joue le rôle de variable d'ajustement. Enfin, le système actuel pâtit d'effets de seuil. Il suffit d'un élève manquant pour fermer une classe ; il en faut bien plus pour en ouvrir Au-delà d'une logique purement comptable, liée à la baisse démographique, nos petites collectivités ont besoin de leurs écoles. Dès lors, monsieur le ministre, comment comptez-vous aider nos communes rurales, tout en prenant en considération le point de vue de leurs maires ? La

Notre ligne directrice est très simple : nous nous adaptons aux réalités démographiques nationales, régionales et locales, tout en accordant une considération particulière à la situation des territoires ruraux.

les territoires ruraux font l'objet d'une attention soutenue. Sur les 33 écoles situées dans les communes les plus rurales, les plus éloignées,

pour vous, madame Couillard, la sauvegarde de la biodiversité et, naturellement, la protection des espaces naturels ; pour vous, monsieur Klein, les très ambitieux 400 000 logements supplémentaires par an pour vous, madame Pannier-Runacher, l'accélération des installations d'énergies renouvelables et de centrales nucléaires ; pour vous, monsieur le garde des sceaux, la construction de nouvelles prisons, ce qui est ; enfin, pour vous, monsieur Béchu, le challenge de répondre aux conclusions de la modérément inspirée Convention citoyenne pour le climat et l'atteinte du fameux « zéro artificialisation nette ». Toutefois, mesdames, messieurs les ministres, vous rendez-vous compte

S'ils ne les exécutent pas toutes, ils sont sanctionnés ! Aucune planification territoriale n'est désormais possible tant les priorités sont nombreuses ! Gouverner, c'est prévoir, c'est choisir ses priorités, c'est donner un cap ; alors, madame la Première ministre- car c'est à vous que je pose cette question je voudrais savoir une chose : dans l'exécution des politiques publiques, quelles sont vos priorités ?

en rappelant précisément la manière dont tout cela doit se faire dans le respect de la planification écologique, tâche qui, par ailleurs, lui a été confiée par le Président de la République. Je vous répondrai d'abord que, parmi ces injonctions contradictoires, il y a ce qui relève du Gouvernement, mais aussi ce que la représentation nationale a pu décider,

par Valérie Létard et Jean-Baptiste Blanc. S'il n'y avait pas à corriger la loi que vous avez votée, nous ne serions pas en train d'avoir cette discussion ici ! Ainsi, il n'était pas prévu, dans la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement,

monsieur le ministre, la réalité est tout autre : les critères que vous appliquez accélèrent la fermeture de classes et d'écoles rurales, avec la suppression de 2 000 postes ! En même temps, le soutien à la ruralité est affiché comme une priorité par les ministres Dominique

Pourquoi, alors que vous poursuivez le dédoublement des classes en zone sensible prioritaire, le monde rural devrait-il payer le tribut d'une approche comptable déséquilibrée ? L'école rurale est une chance pour nos enfants, car elle conjugue proximité et qualité de l'enseignement.

M. Guerriau, votre département du Puy-de-Dôme va perdre 616 élèves à la rentrée 2023. Dès lors, si nous devions

les élèves -va s'améliorer. Nous examinons très attentivement les 491 écoles de votre département, ce qui nous conduit à envisager la fermeture d'une trentaine de classes, mais aussi l'ouverture d'une vingtaine d'autres. En effet, quand nous évoquons les suppressions de classes, nous parlons également d'un solde, c'est-à-dire d'une différence entre les ouvertures et les fermetures.

Monsieur le ministre, vos actions amplifient la fracture territoriale et suscitent la colère des maires et des citoyens

Cessez ce mépris pour les habitants des territoires ruraux, cessez ce sacrifice de la ruralité sur l'autel des quotas et des normes ! Sinon, mesdames, messieurs les ministres, les « Gaulois réfractaires » risquent de se réveiller

Ainsi, certaines villes touristiques font les frais d'une concurrence insupportable entre les logements classiques et les meublés de tourisme. Ne serait-ce qu'en Charente-Maritime, on constate, à Oléron, des abus énormes dénoncés par les élus concernant la collecte et le reversement des taxes de séjour de séjour ; à La Rochelle, le phénomène explose, avec, rien qu'en 2022, plus de 1 700 meublés de tourisme nouvellement déclarés qui évincent autant de travailleurs et d'étudiants en mal de logement. La Rochelle a attaqué le mal à la racine, et ce dès 2019, en soumettant à autorisation préalable la mise sur le marché de meublés de tourisme, grâce à un numéro d'enregistrement unique, et en instaurant, pour les personnes physiques, un dispositif d'autorisation de changement d'usage temporaire des locaux destinés à l'habitation pour des locations de courte durée.

en exigeant des mesures de compensation comme l'obligation de transformer un local en logement à l'année pour chaque logement de tourisme mis sur le marché, ou encore en favorisant la réservation des logements de petite taille par les étudiants ou jeunes actifs vivant seuls. Malheureusement, cette agglomération, comme d'autres, se heurte à un cadre légal et réglementaire dont jouent parfaitement les utilisateurs de plateformes, ainsi qu'à l'appréciation négative par les juridictions de la proportionnalité des mesures mises en oeuvre. Pourtant, avoir un toit pour étudier ou travailler et pouvoir vivre près des siens est le premier élément d'insertion dans la communauté nationale. Alors, monsieur le ministre, quelles mesures vous engagez-vous à proposer, avec le concours de ces collectivités volontaristes et du Parlement ? On ne peut plus laisser la « plateformisation » du logement miner le pacte républicain ! La parole est à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

dit, nous pensons que c'est avec les associations d'élus, en examinant les moyens qu'on pourrait leur donner à l'échelle locale, que l'on tiendra compte de l'hétérogénéité des situations. Là aussi, notre conviction

Depuis des années, les filières avicoles françaises ont oeuvré pour produire des volailles qui répondent aux normes de production, aux exigences du bien-être animal et aux attentes des consommateurs. Ces normes, identifiées par un étiquetage clair et simple, ont permis à la production française de trouver une place sur le marché dans des conditions de concurrence équitables. Mais voilà que la Commission européenne a décidé, à la fin de 2022, d'accorder à tous types d'élevage pleine liberté d'utiliser des labels sans fondement et sans aucun contrôle ! Nous risquons ainsi de voir apparaître des mentions fantaisistes, comme « poulet de plein vent » ou « poulet des champs », qui tromperont le consommateur. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple : quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour sauver ces labels et nos filières avicoles ?

à plusieurs reprises par voie écrite et orale, et lors de conseils européens. Vous avez raison, l'inquiétude règne quant à la réforme des normes de commercialisation qui a été lancée par la Commission européenne et soumise aux États membres, pour avis uniquement. est bien la difficulté, dans le travail que nous avons à accomplir avec la Commission. Dès le début de cette négociation, la France a indiqué son désaccord sur différents points, en particulier sur la révision des dispositions relatives aux mentions valorisantes, réservées ou facultatives, c'est-à-dire aux normes de commercialisation. Vous avez très bien décrit les risques que fait courir ce projet de réforme. Le premier, c'est un risque de tromperie du consommateur,

Vous nous répondez que les éleveurs français doivent monter en gamme pour trouver des marchés avec des marges plus élevées, selon les objectifs de la stratégie ou du. Le bilan de cette approche, c'est que, dans la filière avicole, la ferme France a perdu la bataille face aux importations pour la restauration collective ou les plats préparés. Alors, il nous reste le poulet du dimanche, le poulet labélisé. Mais si vous ne défendez pas ces labels qui nous sont chers, tant pour les producteurs que pour les consommateurs, nous perdrons cette ultime bataille ! Nous constatons tous les jours que les normes et les surtranspositions s'appliquent aux agriculteurs français ; notre administration se développe toujours plus pour contrôler nos productions plutôt que les produits qui sont importés. En conséquence, nos fermes ne sont plus reprises par les jeunes. Vous vous étiez engagé à faire respecter les clauses miroirs ; nous attendons des suites ! Vous acceptez au contraire une nouvelle concurrence déloyale qui se révélera fatale pour nos productions et, probablement, pour les 15 000 emplois ruraux qui dépendent de ces labels. la ferme France brûle, mais nous regardons ailleurs ! La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour le groupe Union Centriste.

Ce texte fixe des objectifs ambitieux d'emploi de l'hydrogène dans l'industrie, ce dont on peut se réjouir, mais il prévoit que cet hydrogène devra être produit à partir d'électricité renouvelable, sans dire un mot de l'électricité produite à partir d'énergie nucléaire. Or, si elle ne peut pas utiliser ses réacteurs nucléaires pour produire de l'hydrogène, la France va avoir beaucoup de mal à atteindre les objectifs européens. L'Union européenne avait déjà tenté sans succès d'exclure le nucléaire de sa taxonomie

en qualifiant cette exclusion de « climaticide » et d'absurde. Nous ne pouvons que vous en féliciter, car le nucléaire est l'énergie la moins carbonée dont nous disposons. Je note par ailleurs que la France est loin d'être le seul État membre frustré par le contenu actuel du texte. Aussi, je voudrais savoir comment se présentent les négociations sur ce sujet.

qui avez adopté hier, à une très large majorité, un projet d'accélération des énergies renouvelables. Je suis d'accord avec vous : il ne faut pas se tromper de combat. Le nôtre, c'est la décarbonation et la défossilisation. Compte tenu de l'ambition de ce combat, nous devons utiliser

décarboné une partie de notre énergie grâce au nucléaire. Il n'est plus question de confondre les moyens- les énergies renouvelables -avec l'objectif final- la décarbonation, la défossilisation.

Les Républicains. Monsieur le ministre de l'éducation nationale, chaque nouvelle évaluation du niveau des élèves

sans aucune considération pour l'école primaire, où se créent les décrochages, et avec pour effet collatéral surprise la suppression de l'enseignement de la technologie. Monsieur le ministre, pouvez-vous révéler à la représentation nationale la méthode de concertation et la stratégie, que j'imagine profonde, vous ayant conduit à prendre une telle décision

Monsieur le ministre, à l'épreuve du grand oral de bac instaurée par votre prédécesseur, votre prestation du jour serait sans doute sévèrement évaluée Aucune thèse dans votre propos, par conséquent pas d'antithèse et encore moins de synthèse ! En réalité, l'éducation nationale prend l'eau de toutes parts et vous écopez à la petite cuillère, dans une forme

Il est grand temps de prendre conscience de l'incurie des concepteurs de nos programmes scolaires, qui fabriquent des générations certes sensibilisées à un tas d'enjeux sociétaux tous plus importants les uns que les autres, mais incapables de calculer un pourcentage et prenant un alexandrin pour un habitant d'Alexandrie. Si vous pensez vraiment qu'il faut changer cela,

et Républicain. Le projet d'union sacrée autour du logement entre les associations et le Gouvernement peine à faire ses preuves.

ces associations ne se contentent pas d'alerter : elles produisent surtout un travail de fond chiffré et documenté- et elles sont les seules à le faire

vous avez raison, le sans-abrisme est une question qui nous préoccupe tous et sur laquelle le Gouvernement agit de manière historique. Hier soir encore, plus de 200 000 places d'hébergement d'urgence étaient ouvertes dans le pays. Ce chiffre n'avait jamais été atteint, jamais été atteint, tous gouvernements confondus. Quelque 5,7 millions d'euros sont dépensés chaque soir pour héberger les plus fragiles- et ce n'est que justice. Le Gouvernement a lancé le plan Logement d'abord

effet, et j'en parlerai dès demain avec l'ensemble de ces maires !

La tribune des vingt maires en question appelle à déployer en urgence un plan stratégique national et transversal qui répondrait à un diagnostic clair et transparent. Le Gouvernement a tout intérêt à produire rapidement celui-ci : cela vous éviterait de contester les seuls chiffres qui existent.

que « les associations sont mal inspirées quand elles tombent dans l'outrance » ; j'ai la modestie et l'humilité de vous dire qu'un gouvernement est mal inspiré quand il tombe dans la suffisance. Bravo ! Ce n'est certainement pas le meilleur moyen de coconstruire. Pour notre part, nous sommes prêts, avec ces

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, en France, de moins en moins d'adultes aspirent à se retrouver devant une classe d'enfants pour les instruire, ou plutôt devrais-je dire de tenter de les instruire Professeur : « le plus beau métier du monde, après le métier de parent », a écrit Charles Péguy. Comme cette affirmation semble d'un autre temps ! Car oui, notre pays vit une crise des vocations sans précédent. Pour certaines matières comme les mathématiques, il y a moins de candidats que de postes à pourvoir.

Dans un contexte de recrutement difficile, plus de 1 600 enseignants ont démissionné en 2021. Le taux de professeurs démissionnaires est même en hausse constante depuis dix ans.

que comptez-vous faire pour réhabiliter enfin la vocation d'enseignant et garantir à nos élèves la transmission d'un savoir sans lequel la promesse républicaine

Madame la ministre déléguée, voilà sept mois que vous êtes en fonction et je souhaite entendre de votre bouche les décisions concrètes que vous avez prises, avec votre ministre de tutelle, pour lutter contre les déserts médicaux. De tous les groupes politiques, de tous les territoires, émanent des rapports successifs, des débats, des questions, des propositions de loi, des amendements sur ce sujet. Par tous les véhicules législatifs possibles, le Sénat attend, propose et exige des décisions efficaces et concrètes pour l'égalité d'accès aux soins de tous les Français, y compris ceux de la ruralité profonde.

Patients abandonnés et maires de France ne peuvent plus supporter cette situation inacceptable et indéfendable. Les décisions courageuses et audacieuses qu'ils attendent dépendent de vous, et non de comités « machin chose » qui consomment du temps et ne ramènent pas la présence médicale dans les territoires. Madame la ministre, que fait le Gouvernement face à ce problème majeur ?

dernier : celui de la refondation de l'ensemble de notre système de santé, qu'il s'agisse de l'hôpital ou de la médecine de ville. À l'hôpital, nous voulons redonner plus de sens, plus de souplesse et plus d'autonomie aux soignants. Cela passe par une meilleure reconnaissance de la pénibilité, mais aussi par une refonte de l'organisation à l'échelle des services ou par une modification de la sortie du tout-T2A (tarification à l'activité). S'agissant de la médecine de ville, nous souhaitons nous inscrire dans une trajectoire à la fois pragmatique, ambitieuse et solidaire.

le débat d'actualité sur le thème : « Quelle réponse européenne aux récentes mesures protectionnistes américaines ? » Je vous rappelle

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat d'actualité sur le thème : « Quelle réponse européenne aux récentes mesures protectionnistes américaines ? » dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l'orateur disposera alors à son tour du droit de répartie, pour une minute. Le temps de réponse du Gouvernement à l'issue du débat est limité à cinq minutes. Madame la secrétaire d'État, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura regagné sa place dans l'hémicycle.

le grand plan d'investissement américain voté l'été dernier retient toute notre attention. Il nous amène à débattre aujourd'hui des réponses que la France et l'Union européenne devraient apporter. L'IRA, ou, est un programme puissant de subventions, mais aussi d'allègements fiscaux de 370 milliards de dollars avec pour objectif de financer la transition écologique et des mesures sociales. Les mesures les plus symboliques sont la création d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique, une subvention pour les fabricants d'éoliennes ou de panneaux solaires utilisant l'acier américain, ou encore une baisse d'impôt pour aider les entreprises dans leur transition énergétique.

Nous ne sommes pas dans un monde de Bisounours, même si nous avons souvent l'impression que l'Union européenne n'en est pas consciente. La première réaction des dirigeants européens a été une levée de boucliers contre ce plan jugé protectionniste accusé les États-Unis de favoriser les investissements sur leur territoire, en visant en particulier et parmi de nombreuses autres mesures l'octroi de certaines subventions délivrées sous condition de relocalisation de la production sur le sol national.

Si nous ne pouvons que soutenir les orientations prises pour répondre au plan d'investissement américain, nous devons également alerter, afin que la Commission européenne fasse preuve de lucidité dans la réorientation des aides allouées ainsi que dans les décisions réglementaires qu'elle pourrait prendre pour développer notre industrie.

inciter le développement industriel sur le sol européen en assurant des avantages fiscaux aux entreprises qui investiront dans le développement d'énergies propres, dans le but final de permettre à l'Union européenne d'assurer sa souveraineté énergétique, donc sa souveraineté économique.

L'onde de choc de la crise énergétique se fait sentir sur le coût de nos importations, avec une hausse de 29 % des importations en valeur, alors que nos exportations, moins sujettes à l'impact de l'énergie, ne progressent que de 18 %. C'est donc plus de 80 % de l'aggravation du déficit qui s'explique par l'augmentation du prix de l'énergie. Même si la France n'a jamais été exemplaire sur sa balance commerciale, ses voisins européens subissent de plein fouet les mêmes effets, avec une baisse de 56 % des exportations par rapport à l'année dernière pour le bon élève allemand. Ce déficit s'explique aussi par la pénurie d'approvisionnement dans certaines matières premières, qui ont pénalisé l'automobile ou l'aéronautique. Cette crise énergétique doit inspirer la politique européenne pour encourager des investissements lourds dans notre industrie, afin que nous soyons en mesure de produire notre énergie décarbonée localement. Il s'agit d'assurer notre souveraineté économique, ne sera garantie que par notre souveraineté énergétique. L'Union européenne a perdu trop de temps à discuter des mois durant afin de savoir si telle ou telle énergie était suffisamment verte pour être subventionnée. Je pense bien sûr aux débats qui ont eu lieu autour du nucléaire. Le plan d'investissement des États-Unis favorise fortement la relocalisation de la production sur leur territoire. L'IRA offre des atouts de compétition, qui, couplés à un prix de l'énergie très faible dans ce pays, font courir des risques à notre industrie. La Commission européenne a communiqué le 1 février dernier que des subventions équivalentes à celles que proposent les États-Unis seront autorisées. Les États membres pourront égaler le montant de l'aide qu'une entreprise européenne se verrait offrir par un pays tiers, comme les États-Unis. un signe encourageant, qui ne permettra sans doute pas à tous les pays européens de réagir de la même manière : tous n'en ont pas les moyens. Annoncer l'octroi de subventions ou d'avantages fiscaux est un premier pas, mais cela devra impérativement être accompagné d'une débureaucratisation de Bruxelles en assurant des obtentions de subventions restreints. Les États-Unis sont très rapides, un peu comme nous l'avons été au moment de la crise du covid-19. Je crains qu'en France et en Europe les entreprises ne soient découragées par la bureaucratie européenne et par des versements de subventions qui prennent plusieurs mois, quelquefois plusieurs années. Au-delà des délais administratifs, la réponse de l'Union européenne doit s'inscrire dans le temps long. Nous avons une fâcheuse tendance à modifier tous les six mois les plans européens pour répondre à telle ou telle urgence. Ce plan doit s'inscrire dans la continuité afin de ne pas décourager les entreprises. Je pense également à notre agriculture, qui a subi de nombreuses réglementations ces dernières années, poussant nos agriculteurs à développer l'agriculture biologique avec le succès mitigé que nous connaissons. Il y a encore quelques jours, la Cour de justice de l'Union européenne a définitivement barré la voie à l'utilisation de néonicotinoïdes, pour seulement deux pays, la France et la Belgique. Il est impératif de s'assurer que ces règles s'appliquent sur l'ensemble des produits que nous importons, afin que nos agriculteurs ne se retrouvent pas face à une concurrence déloyale. La confiance de nos concitoyens dans l'Union européenne est de plus en plus fragile, face à des règles fermes pour nos producteurs, mais faibles quant à leur application à des produits importés.

Madame la secrétaire d'État, quelles réponses l'Union européenne peut-elle apporter à ce plan d'investissement américain ? La technostructure européenne ou française sera-t-elle capable d'apporter une réponse rapide avec des déblocages immédiats des fonds, comme savent le faire les Américains ? ? L'Union européenne est-elle prête à instaurer des normes barrières afin de réduire la pénétration de son marché par les produits américains ou chinois ? L'Europe va-t-elle enfin se réveiller face à la concurrence internationale, sachant qu'elle est beaucoup plus handicapée notamment par les conséquences du conflit ukrainien ?

globale. De nouveaux instruments de défense commerciale ont notamment été développés pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne ; je pense en particulier à l'instrument antisubventions qui nous permettra

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, dans le climat de contestation générale du multilatéralisme, les règles du commerce mondial n'échappent pas à la tendance. De l'de Donald Trump aux aides d'État de Joe Biden, les États-Unis semblent s'en affranchir de plus en plus.

Au travers de ce fameux IRA, l'Oncle Sam s'apprête à déverser 369 milliards de dollars de subventions aux entreprises qui investiraient dans la transition verte sur le sol national. La bonne nouvelle, vous l'indiquez, madame la secrétaire d'État, c'est que les États-Unis confirment avec ce plan qu'ils ont pris la mesure de l'urgence climatique. La mauvaise, c'est qu'ils nous ont vendu pendant des décennies le concept d'une « mondialisation heureuse », pour aujourd'hui jouer leur propre partition de relocalisation. Comme vous le savez, mes chers collèges, l'IRA inquiète nos entreprises, nos territoires et les pouvoirs publics. Après l'épreuve de la pandémie qui a affecté notre économie, puis celle de la guerre qui renchérit le prix de l'énergie, le projet américain pourrait en effet fragiliser un peu plus le tissu industriel européen. Depuis l'annonce américaine au mois d'août dernier, on entend que Saint-Gobain voudrait s'agrandir en Californie, que Volkswagen augmenterait ses capacités de production de l'autre côté de l'Atlantique, tout comme le fabricant suédois de batteries Northvolt. Madame la secrétaire d'État, avez-vous quelques éléments précis concernant les groupes français qui seraient tentés par le nouveau rêve américain ? En attendant, comme nous y invite ce débat, il nous faut nous interroger sur les réponses que l'Union européenne peut apporter à ces mesures protectionnistes. Le Conseil européen du mois de décembre dernier a bien souligné « la nécessité d'une réponse coordonnée pour renforcer la résilience économique de l'Europe et sa compétitivité sur le plan mondial, tout en préservant l'intégrité du marché unique ». qui est de la réponse coordonnée, on peut avoir une inquiétude au regard des positions divergentes de certains États membres en fonction des propositions avancées par Bruxelles. Cependant, je me réjouis que Paris et Berlin s'entendent sur l'assouplissement des aides d'État liées à la transition écologique, ainsi que sur la simplification des règles d'installation des usines. Le groupe RDSE est en tout cas favorable à cette première réponse. Je n'oublie pas une difficulté intrinsèque à l'Union européenne, à savoir l'existence de règles régissant le marché unique qui compliquent l'octroi de subventions aux entreprises. Sur ce point, l'Union européenne ne doit pas être dogmatique, sous peine de rester la variable d'ajustement dans un monde dérégulé.

Je souligne toutefois qu'il ne s'agit pas d'entrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis, certainement pas dans le contexte de la guerre en Ukraine qui nécessite un lien fort entre alliés. Une autre réponse pourrait consister en la création d'un fonds de souveraineté européen. RDSE, attaché à la cohésion de l'Europe et à la solidarité entre États membres, telle qu'elle s'est exercée au travers du plan de relance, est ouvert à cette idée. Je rappelle que ce fonds suscite l'intérêt de la Banque publique d'investissement. On peut relever que Bpifrance a su jouer son rôle dans la mise en oeuvre du plan Juncker. Madame la secrétaire d'État, plus globalement, ce débat pose la question de l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Bien qu'il soit clair que l'Union européenne ne sera jamais autosuffisante, la réponse au plan américain doit être celle de la reconstitution d'une industrie compétitive irriguant tous les territoires.

l'investissement dans les secteurs industriels et de service nécessaires à cette transition, elle ne peut qu'être saluée. L'inquiétude provient cependant du volume considérable des subventions qui vont être consenties par les autorités américaines- près de 370 milliards de dollars -et, surtout, du fait que l'accès à ces financements ou avantages fiscaux sera réservé aux productions localisées sur le territoire des États-Unis. Combiné au coût bien moindre de l'énergie et à d'autres facteurs avantageant déjà les États-Unis par rapport à l'Union européenne, ce plan de soutien massif risque de créer un effet d'attraction quasi irrésistible pour la localisation ou la relocalisation d'investissements européens dans ces secteurs d'avenir aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Face à ce danger de concurrence déloyale, l'Union européenne ne peut pas rester sans réaction. Elle a exprimé sa préoccupation à ce sujet au plus haut niveau et à plusieurs reprises, mais elle se trouve véritablement mise devant le fait accompli, puisque, comme je l'ai signalé, la loi IRA est déjà entrée en vigueur. L'Union européenne et les représentants de la France doivent donc réagir rapidement, en mettant en place tous les éléments d'une réponse européenne appropriée. Avec leurs clauses de localisation obligatoire des productions subventionnées sur le territoire des États-Unis, les aides américaines enfreignent clairement les disciplines de l'OMC. Les contester à Genève pourrait cependant se révéler contre-productif, dans la mesure où le mécanisme de règlement des différends de l'OMC est devenu largement inopérant du fait de la paralysie de l'organe d'appel et qu'il est clair que les États-Unis n'ont aucune intention de se plier à d'éventuelles recommandations formulées dans ce cadre. Amener l'administration américaine à revoir son dispositif ou à aménager certaines exceptions en faveur de l'Union européenne, comme celles qui sont prévues pour le Canada et le Mexique, est mission impossible. Elle a clairement fait comprendre à ses interlocuteurs européens, y compris le Président de la République lors de sa récente visite d'État à Washington, qu'elle n'était nullement disposée à le faire. Il reste donc aux Européens à trouver par eux-mêmes des remèdes adéquats au danger auquel ils se trouvent ainsi confrontés. Une piste envisagée, en direction de laquelle des dispositions ont déjà été prises, consiste à assouplir ou suspendre une nouvelle fois les règles européennes concernant les aides d'État pour autoriser les États membres qui le souhaitent et qui le peuvent à soutenir les activités concernées sur leur territoire. L'inconvénient de cette approche est double : elle favorise les seuls États qui peuvent se le permettre financièrement- la France en fait-elle encore partie ? j'en doute -et elle remet en question le principe de concurrence loyale, le, sur lequel est fondé le bon fonctionnement du marché unique européen. Une autre piste, fortement privilégiée par la France, mais loin de faire l'unanimité chez ses partenaires, consisterait à déployer un plan européen similaire au plan américain et d'un montant suffisant pour inciter les opérateurs des secteurs concernés à privilégier les investissements en Europe. Comment mobiliser autant d'argent à l'échelon européen- on parle de 300 à 350 milliards d'euros -, alors que l'Union européenne vient à peine de mettre en oeuvre un plan de relance post-covid de 750 milliards d'euros. Une partie de ce plan existant pourrait sans doute être réorientée vers un tel « fonds européen de souveraineté », comme l'envisage la Commission européenne, mais cela ne suffira certainement pas à faire la différence. Cette initiative américaine met donc l'Union européenne dans un embarras dont elle aura bien du mal à se tirer, ce qui m'inspire les réflexions suivantes. Les États-Unis font, une fois de plus, preuve d'un égoïsme sacré en menant une politique décomplexée d', qui ne tient qui ne tient absolument pas compte des retombées négatives de leurs initiatives pour leurs partenaires traditionnels. Ils restent les princes du protectionnisme. Ceux qui croyaient naïvement que l'arrivée au pouvoir d'une administration démocrate à l'issue du mandat de Donald Trump conduirait nécessairement à une amélioration significative des relations transatlantiques en sont pour leurs frais. Le style a changé, la rhétorique utilisée aussi, mais aucune concession réelle n'est faite sur le terrain des intérêts économiques et commerciaux. On aurait pu penser que le contexte géopolitique conduirait les États-Unis à mieux soigner leurs relations avec leurs alliés afin de ne pas ouvrir de brèches trop visibles dans la coalition occidentale. Malheureusement, il n'en est rien et ces considérations de politique étrangère semblent peser assez peu par rapport aux objectifs de politique intérieure américaine que l'administration Biden cherche à atteindre Ce constat ne peut en tout cas qu'inciter l'Europe et la France à faire de l'autonomie stratégique dans tous les domaines- énergie, agriculture, industrie, recherche, défense -l'un de leurs objectifs les plus fondamentaux et à tout mettre en oeuvre pour l'atteindre dès que possible. Le général de Gaulle avait eu l'intuition de cette impérieuse exigence dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Elle a malheureusement été perdue de vue pendant des décennies, dans un contexte de mondialisation débridée. Il est grand temps, selon moi, qu'elle revienne au premier plan dans les préoccupations de nos décideurs, dont vous êtes, madame la secrétaire d'État.

la réciprocité sur les marchés publics et l'instrument antisubventions. Enfin, lors de son voyage aux États-Unis, Bruno Le Maire a obtenu une alliance sur les matériaux critiques, pour que nous nous fournissions de façon diversifiée et en coopération avec les États-Unis. avec les États-Unis. Le différentiel de compétitivité est principalement dû au différentiel de prix de l'énergie dont nous souffrons plus

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la guerre commerciale que l'Union européenne et les États-Unis se livrent est inversement proportionnelle à leur relation en tant qu'alliés. Ces deux grandes puissances, aux multiples combats communs, sont celles qui s'affrontent le plus dans le domaine commercial

Régulièrement, la presse titre sur une nouvelle guerre commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Cela ne date pas d'hier ; cela ne date pas non plus de la présidence Trump. En effet, après quatre années de trumpisme, les Européens promettaient de développer enfin leur souveraineté pour ne plus avoir à subir les choix politiques américains.

Bien naïf celui qui pensait le contraire ! Réarmer nos souverainetés est un projet de long terme, indispensable à bien des égards. La crise du virus chinois,

La crise énergétique actuelle risque fortement de déboucher sur un choc de compétitivité et une crise plus durable en Europe, ce risque étant encore plus élevé du fait des dernières mesures protectionnistes prises par les États-Unis.

en développant l'hydrogène vert, les batteries, le solaire, l'éolien, la rénovation énergétique des bâtiments, les véhicules électriques ... Cette énumération a un goût de déjà-vu de notre côté de l'Atlantique, bien plus avancé sur ces sujets.

qu'on osait à peine murmurer en une réalité solide et concrète. Aujourd'hui, être européen, c'est être conscient de la nécessité d'agir ensemble. Nous devons nous protéger en toute indépendance.

Le sommet extraordinaire qui se tiendra demain et après-demain nous y invite. Après les derniers Conseils européens, nous sommes inquiets quant à notre capacité à trouver une solution commune. Tout en saluant la feuille de route pour le renforcement de la politique industrielle, je relève

de retrouver notre souveraineté. Ce n'est pas seulement la guerre économique ou la réponse européenne au protectionnisme américain qui se joue là, même si nous espérons cette réponse puissante. Les enjeux sont plus larges et ne doivent pas faire oublier d'autres tensions. La bataille que nous devons mener est celle des idées et celle d'un modèle. Affirmons haut et fort que nous sommes, avant tout, des Européens ! La parole

ont conçu la contre-offensive et transmis leur contribution à la Commission européenne. Mme von der Leyen a ensuite dévoilé, à Davos, ses mesures face à l'IRA. Cette évolution renvoie à ce que nous, écologistes, prônons : un protectionnisme vert européen. Cela consiste, d'abord, à mettre en cohérence les règles de notre marché intérieur et nos importations. Sur le plus long terme, il s'agit de réindustrialiser l'Europe pour lui permettre d'être plus autonome, plus souveraine, en cessant d'avoir pour boussole le productivisme mondialisé.

assumer notre place de premier marché au monde et affirmer que l'accès à ce marché impose le respect de critères fondés sur nos valeurs. On ne peut plus polluer impunément avec des biens vendus à des prix qui ne reflètent pas du tout les externalités négatives causées En réponse à l'IRA, la Commission européenne a mis en avant des objectifs de réindustrialisation par le biais d'allégements de cotisations, notamment pour le déploiement de nouvelles technologies. Elle souhaite aussi autoriser davantage d'aides d'État et de crédits d'impôt pour les technologies vertes. Toutefois, un levier majeur manque : un. Proposé par

14 % du PIB européen. C'est de l'argent qui existe déjà et un levier de transformation déterminant. Utiliser les marchés publics, c'est offrir une protection aux Européens effrayés par la mondialisation, le chômage et ce qu'implique de mutations la transition écologique. Mais c'est surtout un levier, qui peut être compatible avec les règles de l'OMC, pour créer des emplois durables et décarboner nos économies.

Le candidat Emmanuel Macron l'avait proposé en 2017 dans son programme, mais cet engagement a été abandonné en faveur d'un libéralisme de la compétition de tous contre tous. Seule l'Europe ouvre ainsi à tous les vents ses marchés publics. Les autres savent les protéger. Nous avons enfin convenu d'une taxe carbone à la frontière : continuons sur cette lancée ! Nous avons décidé de fermer notre marché à des produits issus de la déforestation. Notre impact est mondial, palpable, mais trop lent. Les États-Unis, eux, décident d'abord et discutaillent après. Sur le photovoltaïque, nous avons été timorés. Nous avons mis tellement de temps à négocier pour tenter de parer la menace chinoise que nous avons raté le train. C'est une bataille politique, et non pas technique.

pragmatiques : les délocalisations ont fragilisé des territoires et détruit des emplois. Un projet écologique et social crédible, c'est la possibilité de consommer des produits venant de chez nous et de pays qui respectent les normes en vigueur chez nous. C'est pourquoi la France devrait insister lors du Conseil pour obtenir enfin les fameuses clauses miroirs sur l'agriculture qu'elle entendait faire adopter sous sa présidence. On ne les trouve pas dans l'accord avec le Mercosur, qui n'est que mondialisation de la malbouffe et de la souffrance animale et qui signe la disparition de nombre de nos paysans. La France a malheureusement l'habitude de faire des propositions intéressantes, de les afficher, puis de renoncer lors des négociations. Pour le, elle a appliqué le même mode opératoire : on propose, puis on baisse les bras au premier froncement de sourcils. de sourcils. Il faut prendre son bâton de pèlerin, créer des alliances, trouver une majorité au Conseil. Ce ne sera pas facile, certes, mais en quelques années, nous avons obtenu des avancées qu'on pensait impossibles taxe sur les superprofits énergétiques, interdiction des importations issues du travail forcé, impôts sur les sociétés, devoir de vigilance, taxe carbone aux frontières ... Les écologistes saluent ces avancées. L'Europe se fortifiera en les approfondissant. La parole est

mesures miroirs. La commande publique représente en effet 14 % du PIB européen. C'est un levier extrêmement important pour la stratégie du, par laquelle nous travaillons à l'inclusion effective de critères qualitatifs dans la commande publique et les dispositifs de soutien à la demande, le tout dans le respect des principes de non-discrimination et de libre accès à la commande publique. L'objectif est d'ouvrir prioritairement les marchés publics à des entreprises qui respectent pleinement les normes sociales et environnementales européennes.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, il y a deux semaines, en première lecture, nous adoptions ici même le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction

salon HyVolution 2023, que j'ai eu plaisir à visiter, la ministre de la transition énergétique dévoilait les nouveaux lauréats de l'appel à projets « Écosystèmes territoriaux hydrogène Depuis vendredi, les élus locaux peuvent demander le financement de leurs projets durables dans le cadre du fonds vert, plus de 3 milliards d'euros de crédits et de prêts étant mobilisés Chers collègues, ces trois actions françaises témoignent de notre volonté d'aller plus loin, et encore plus vite, pour atteindre les objectifs fixés pour 2030 en matière de réduction d'émissions carbone. En Europe, le cap est également fixé : zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050. C'est demain ! Pour atteindre cet objectif, plusieurs leviers ont été proposés par nos instances européennes : la feuille de route « Ajustement à l'objectif 55 » ; un plan pour aider à réparer les dommages économiques et sociaux immédiats causés par la pandémie,, doté de 725 milliards d'euros, dont 40 % pour la transition écologique ; enfin,, un plan de bataille de l'Union européenne pour gagner en indépendance énergétique, qui permettra notamment de développer les filières de recyclage des énergies renouvelables. Ce sont autant de leviers pour guérir, prévenir, anticiper, refonder, innover. À l'heure où nous parlons, le Conseil européen discute d'un nouveau plan industriel, un Pacte vert pour l'Europe, visant à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne à zéro émission nette et à soutenir une transition rapide vers la neutralité climatique. Il a été présenté la semaine dernière par la présidente von der Leyen. À l'issue de ces échanges, une proposition juridique devrait aboutir d'ici à la mi-mars et pour le temps long. Nous abusons parfois de l'hyperbole, mais le fait est que nous sommes véritablement à un tournant historique.

Si nous nous réjouissons que les grandes économies intensifient leurs investissements dans l'industrie à zéro émission nette, cela ne peut se faire au détriment d'une concurrence équitable et transparente. Alors que nous cherchons un cadre réglementaire européen approprié pour nos industries, plus simple, plus efficace et prévisible, nous ne pouvons pas tolérer d'éventuelles distorsions de concurrence. C'est pourquoi les ministres de l'économie français et allemand se sont déplacés hier auprès de leurs homologues américains. Nous devons défendre notre industrie verte européenne et lever les freins. Cela passe par le volet réglementaire, par la simplification et l'accélération de la procédure des projets importants d'intérêt européen commun (Piiec) ; l'adaptation des règles en matière d'aides d'État pour autoriser le soutien ciblé à certains secteurs clés de la transition verte,

pourraient être utilisés à cet effet. Enfin, en tant qu'Européens, nous devons mettre un point d'honneur à former et à recruter davantage dans les métiers de demain. Je pense aux ingénieurs, techniciens, soudeurs dans le secteur des énergies renouvelables, du nucléaire ou de la fabrication des composants électroniques, dont nos industries manquent cruellement. En plus de ces réponses européennes, il nous faut poursuivre les négociations avec nos partenaires, notamment les États-Unis. Nous devons obtenir des exemptions pour les entreprises européennes dans le cadre des enceintes consacrées à ces questions et rétablir des conditions de concurrence équitables. Madame la secrétaire d'État, chers collègues, il n'y a pas de doutes possibles : dans ce contexte, l'Europe est évidemment

de prêts et 20 milliards de dons aux pays européens. En complément, nous demandons aussi à la Banque européenne d'investissement, qui se dit banque du climat, de se mobiliser et de réfléchir

La parole est à M. Didier Marie. Après l'urgence de la crise sanitaire, après les épreuves imposées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences sur l'ensemble de l'Europe, la vague protectionniste des grandes puissances est un nouveau défi de taille pour l'Union européenne et son marché unique. L'adoption de l'IRA par le Congrès américain et le déblocage de quelque 370 milliards de dollars pour prendre le virage écologique va doper l'industrie et la consommation aux Si cette décision de l'administration Biden est à saluer pour ce qu'elle représente en termes de réponses au défi du dérèglement climatique et d'amélioration des conditions de vie des ouvriers, elle porte en germe le risque de délocalisations massives d'entreprises européennes, confrontées à une énergie chère et à un encadrement strict des subventions. Il convient, dans ce contexte, de ne pas négliger l'autre grande puissance, la Chine, qui a elle aussi pris le virage des technologies vertes à grand renfort de subventions d'État et de travail à bas coût. Face à ce virage historique et à ce retour du protectionnisme, l'Union européenne et l'ensemble des États membres se doivent de réagir. Ce changement de paradigme doit pousser l'Union européenne à être plus ambitieuse pour engager une réelle transition écologique. Le débat d'actualité de ce jour est donc le bienvenu pour évoquer ensemble les positions à tenir. L'Union européenne ne part pas de zéro, tant s'en faut, même si les mesures déjà prises pour la compétitivité et la préservation de nos intérêts stratégiques l'ont trop souvent été en réaction aux crises et non par anticipation, ce que l'on peut regretter. Dans le cadre des mesures de défense commerciale, la réglementation antidumping modernisée en 2018, le filtrage des investissements de pays étrangers ou encore les mesures de sauvegarde, sont déjà actés. Le règlement relatif aux subventions étrangères, entré en vigueur au début du mois de janvier, le et l'instrument du marché unique pour les situations d'urgence, à venir, sont également des outils pertinents pour l'autonomie stratégique, qu'il conviendra d'utiliser sans remords. La présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, a présenté le 1 février les contours d'un plan industriel, dit Pacte vert. C'est une bonne nouvelle, et les instances européennes ne doivent pas hésiter à avoir recours à des dispositifs innovants : nous ne devons avoir aucun tabou.

une loi sur les matières premières critiques et la tant attendue réforme du marché européen de l'électricité. Si ces propositions semblent aller dans le bon sens, nous suivrons avec attention la réforme du marché de l'électricité, celui-ci soit enfin porté par une logique d'intérêt général et adapté à notre mix énergétique et qu'il protège efficacement les entreprises et les citoyens européens. Deuxièmement, la présidente von der Leyen a annoncé un accès plus rapide à des financements, essentiellement grâce à un assouplissement de l'encadrement du régime des aides d'État,

Toutefois, après les premières annonces, bienvenues, de la présidente de la Commission lors du forum de Davos, la Commission semble tergiverser, sous la pression des intérêts contradictoires de certains États membres. Madame la secrétaire d'État, la France doit s'engager avec force et volonté dans les négociations européennes. Permettez-moi de formuler quelques interrogations. Quelle est à ce stade la définition des « technologies propres » ? Quels secteurs seront précisément concernés par ce plan ?

Enfin, la simplification administrative annoncée par la Commission ne doit pas se transformer en une dérégulation à outrance, où la recherche de compétitivité se traduirait par un contournement permanent des normes sociales et environnementales. L'absence d'un pilier social dans ce plan est également préjudiciable, car le sujet de la construction de l'Europe sociale ne peut pas être relégué au second plan. Nous avons, madame la secrétaire d'État, suivi et entendu les nombreuses déclarations du Président de la République et du ministre de l'économie

Il serait intéressant à cet égard que vous nous donniez de plus amples informations sur les résultats obtenus par Bruno Le Maire et son homologue allemand, Robert Habeck, lors de leur déplacement hier à Washington, notamment sur les potentiels accords de réciprocité et les actes de coopération, comme nous avons pu en obtenir sur les semi-conducteurs. Toutefois, je pense qu'il ne faut pas excessivement miser sur l'assouplissement des positions américaines, compte tenu du contexte interne aux États-Unis. Le président Biden n'a obtenu que difficilement l'accord du Congrès et, même s'il le souhaitait, ce qui n'a rien d'évident, il lui serait difficile d'en modifier les termes. Cependant, la Commission européenne pourrait utilement s'inspirer de ses ambitions en faveur de la transition écologique et des intérêts des travailleurs américains. L'Europe doit réagir, non pas par des mesures de rétorsion- nous n'avons aucun intérêt à une guerre commerciale -, mais en mettant en oeuvre un plan ambitieux pour ne pas être marginalisée dans la compétition économique mondiale.

Alors que les États-Unis ont fait le choix de mettre 370 milliards de dollars sur la table, jusqu'où la Commission et le Conseil sont-ils prêts à aller ? Des divergences sont déjà apparues lors de la réunion du Comité des représentants permanents

En complément de la taxation sur les bénéfices des multinationales à hauteur de 15 %, qui entrera en vigueur le 31 décembre 2023, d'autres solutions existent : l'extension du marché carbone européen, la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou encore la création d'une nouvelle taxe sur les transactions financières.

Dans ce cadre, la Banque européenne d'investissement devra jouer pleinement son rôle et devenir le prêteur le plus vert au monde. Le deuxième enjeu est d'éviter l'entrée en guerre commerciale et l'enlisement dans une spirale protectionniste. L'Union européenne doit se dégager de l'étau de l'affrontement sino-américain et poursuive sa stratégie d'ouverture au reste du monde, en développant les accords commerciaux tout en faisant preuve d'une vigilance et d'une exigence extrêmes s'agissant Le troisième enjeu porte sur le développement des compétences- objectif européen de l'année 2023 -, indispensable pour qualifier les salariés des secteurs d'avenir et réussir les transitions numérique et écologique. La reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles évoquée par la Commission est importante pour faciliter les mobilités internes des travailleurs, mais elle devra s'accompagner d'échanges sur la création d'emplois de qualité et sur la dignité au travail. Pour conclure, la réponse aux mesures protectionnistes des États-Unis, qui ont délibérément contourné les règles de l'Organisation mondiale du commerce, devra être d'ampleur, globale et ambitieuse. Il nous faut éviter une guerre commerciale avec les États-Unis et négocier tout ce qui peut l'être,

ont d'abord convenu avec Washington de la nécessité, pour l'application de l'IRA, d'élargir les exemptions au plus grand nombre de composants européens possible, que ce soit pour les véhicules électriques ou les matériaux critiques. Un groupe de travail sur les matériaux critique sera mis en place

d'un enjeu capital pour l'avenir de nos industries, pour notre agriculture, pour l'emploi et pour le développement des territoires. Les États-Unis, qui n'ont jamais été avares de mesures protectionnistes, engagent à présent 370 milliards de dollars dans leur loi de réduction de l'inflation, auxquels il faut ajouter les 52 milliards de dollars de subventions directes issues de leur. Leur objectif est de développer leur industrie et leurs technologies vertes, sans concertation avec leurs partenaires, notamment l'Union européenne.

Les dirigeants nord-américains ont donc décidé d'amplifier la guerre économique pour regagner des parts de marché mondiales et stimuler leur croissance. Cet engagement pour le climat ne doit pas servir de prétexte pour affaiblir l'industrie et l'agriculture européennes.

avec l'offensive guerrière de Poutine et que l'environnement est un prétexte pour dominer de nombreux secteurs industriels, le tout sur fond du recul prévisible des pays occidentaux dans la production des richesses mondiales.

Ils cherchent à rendre leur pays attractif pour les entreprises d'avenir, celles qui mettront en place les technologies performantes de demain, en captant pour leurs sociétés multinationales des savoir-faire, des brevets, des compétences et des entreprises. Ils le font, évidemment, en contradiction avec les théories du libre-échange, qu'ils prônent notamment au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Ils le font dans le cadre de la guerre, qui les sert si bien pour affaiblir les industries automobiles allemande et française, mais aussi une multitude d'autres activités, qu'ils réimplantent dans une Europe qu'ils avaient quelque peu délaissée. Ils le font en utilisant l'arme supplémentaire dont ils disposent : leur monnaie, la référence dans les échanges internationaux.

Face à un tel risque de perte de souveraineté économique pour l'Union européenne, nous ne pouvons rester les bras ballants. Nous n'avons aucun intérêt à nous asseoir, encore, dans le fourgon américain. Déjà, on parle de plus en plus, dans les milieux d'affaires, de délocaliser une part de nos productions aux États-Unis et au Canada pour profiter d'une énergie moins chère. Ce serait une nouvelle catastrophe pour l'emploi. Nous pouvons pourtant nous défendre en consolidant nos marchés publics, qui représentent de 14 % à 19 % du produit

De même, lorsque des secteurs entiers sont à ce point menacés, il est possible de déclencher la clause de sauvegarde. Autrement dit, nous n'avons aucun intérêt à adopter une attitude suiviste à l'égard des États-Unis. Il nous faut au contraire faire entendre une voix autonome, pour obtenir un cessez-le-feu et parvenir à la paix en Ukraine. Chacun comprend bien que l'alignement sur la stratégie militaire américaine empêche l'Union européenne, et surtout la France, de défendre ses intérêts stratégiques. Or nous devrions avoir l'audace de bâtir des consortiums européens publics dans des secteurs comme le numérique, l'hydrogène vert ou encore l'énergie solaire, en favorisant des coopérations dans l'industrie automobile de demain, le transport maritime ou aérien. Nous devrions avoir l'audace de réviser le marché unique de l'énergie, qui est un frein au développement. Enfin, nous devrions avoir l'audace de modifier les règles budgétaires européennes afin de favoriser les investissements du futur. De ce point de vue, un fonds de développement européen offrant des crédits à taux nul serait utile et efficace. Veuillez conclure, mon cher collègue ! Les aides d'État, comme les crédits européens, doivent être conditionnées aux investissements verts et à la création d'emplois. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, voilà trente ans, le sommet de la Terre à Rio donnait le coup d'envoi de l'action mondiale pour le climat.

défi, à la fois économique et conceptuel : économique tout d'abord, car l'ambition portée par l'IRA n'est pas seulement climatique ; elle est aussi, et peut-être avant tout, industrielle. Certes, les 370 milliards de dollars de ce plan de soutien doivent permettre aux États-Unis de réduire leurs émissions de 42 % d'ici à 2030, mais ils doivent surtout assurer l'émergence d'une industrie verte puissante, assise sur des chaînes d'approvisionnement relocalisées et capable de prendre la tête de la course mondiale aux technologies propres. Avec ses exigences de localisation du contenu et de l'assemblage des produits subventionnés, l'IRA envoie un message extrêmement clair : les fonds publics américains ne profiteront qu'au. Ce faisant, Ce faisant, les États-Unis s'offrent un avantage comparatif considérable dans l'un des rares domaines industriels, celui des technologies bas-carbone, dans lequel l'Europe peut se prévaloir d'une avance certaine. Ce domaine sera, rappelons-le, la clé de voûte de l'industrie mondiale de demain. Il transformera des secteurs entiers aussi rapidement qu'il créera de nouveaux marchés. Au moment où nos industries subissent une explosion des prix de l'énergie, qui épargne leurs concurrentes américaines, l'IRA pourrait bien leur porter Alors que les écarts de compétitivité ne cessent de se creuser, le risque de délocalisation vers les États-Unis devient en effet systémique. Les décisions d'investissement annoncées ces derniers mois par plusieurs grands groupes américains comme européens attestent d'ailleurs de la réalité de cette menace. Selon la Première ministre, le plan américain pourrait, à court terme, faire perdre 10 milliards d'euros d'investissement à la France et compromettre quelque 10 000 créations d'emploi.

Tout d'abord, parce que là où l'Europe, avec le, conçoit sa politique environnementale en imposant des standards et des normes, les États-Unis, avec l'IRA, mettent en oeuvre une politique industrielle offensive. Ensuite, parce que les Américains abordent le défi de la transition écologique comme ils l'ont toujours fait : avec pour seule boussole la défense de leurs intérêts économiques. Ne nous leurrons pas : dans cette perspective, l'Europe n'entre à aucun moment en ligne de compte.

Nous ne devrions toutefois pas être surpris que les Américains usent d'un protectionnisme assumé. Ils le pratiquent, au gré de leurs intérêts, depuis au moins un siècle. N'oublions pas que le est en vigueur depuis 1933 depuis 1933 ! L'Europe doit aujourd'hui regarder toutes ces réalités en face et réagir. Bien sûr, les discussions entamées avec les autorités américaines sur l'IRA peuvent être utilement poursuivies. Il semblerait même qu'elles aient produit de premiers résultats encourageants. Tant mieux, mais il semble clair que si des ajustements sont obtenus,

C'est donc avant tout par ses propres moyens que l'Europe doit répliquer aux distorsions de concurrence. Une chose est sûre : pour répondre aux Américains, pour réussir sa transition verte et numérique et pour rester une terre de production, il faudra qu'elle soit en capacité d'attirer des investissements et donc d'envoyer les bons signaux. L'annonce d'aides d'État plus simples, plus rapides et ciblées sur l'ensemble de la chaîne de valeur est ainsi une inflexion de doctrine qui va dans le bon sens et qui pourrait d'ailleurs être étendue à d'autres pans de la politique de concurrence. Attention toutefois à ne pas déstabiliser le marché unique par des volumes de subventions qui seraient trop disparates selon les États membres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Commission proposera de créer en complément un fonds de souveraineté européen. Selon Thierry Breton, 350 milliards d'euros devraient être mobilisés pour soutenir les projets industriels structurants. L'idée est évidemment séduisante, mais la question de son financement reste entière, en particulier s'il devait être proposé d'émettre une nouvelle dette commune. Les oppositions de principe seraient alors nombreuses et nourries par le fait que, à ce jour, l'Europe ne sait toujours pas précisément comment elle remboursera son plan de relance. D'autres pistes de réflexion, plus techniques, sont également sur la table. On le voit néanmoins, l'Union cherche encore le bon calibrage pour faire face à l'IRA et, plus largement, pour bâtir enfin une politique industrielle commune efficace. Elle devra pourtant faire vite. À cet égard, le sommet européen des deux prochains jours ne devra pas déboucher sur des mesures. Il doit surtout être l'occasion pour les Européens de pousser plus loin leur réflexion, car, pour donner un nouvel élan à notre industrie, d'autres leviers structurels doivent être actionnés. Je pense notamment à l'environnement réglementaire des entreprises, qui reste trop complexe et contraignant, au développement des compétences, qui font trop souvent défaut aux industries et, bien sûr, aux prix de l'énergie, pour lesquels nous attendons encore et toujours une réforme efficace du marché européen de l'électricité. Avant tout, l'Union européenne doit adapter son logiciel de pensée. Face aux grandes mutations de l'économie mondiale, face à la déliquescence du multilatéralisme commercial, face aux stratégies développées par les États-Unis et par tant d'autres, à commencer par la Chine, pour protéger et favoriser leurs entreprises, notre continent ne peut rester sans réaction. Il devra, tôt ou tard, se résoudre à jouer à armes égales avec ses concurrents. Quelques avancées ont eu lieu pour établir un cadre stratégique de soutien au développement industriel, par exemple la mise en oeuvre des projets importants d'intérêt européen commun. Mais, pour que les leaders industriels apparaissent ou se maintiennent dans les secteurs stratégiques de demain, l'Europe devra faire de la réciprocité le maître mot de sa stratégie économique et commerciale. Dès lors, elle ne doit plus s'interdire de renouer avec le concept de préférence communautaire. À l'instar de ce que prévoit l'IRA, l'Union et ses États doivent pouvoir imposer dans leurs programmes de subventions des exigences en termes de localisation des approvisionnements et de production. les États de l'Union doivent pouvoir réserver une part de leur commande publique aux entreprises produisant en Europe. À rebours des politiques menées ces dernières décennies, c'est donc une véritable stratégie du qu'il faut développer pour conforter la base industrielle de l'Union. En renforçant l'arsenal de ses outils de défense commerciale, en adoptant un instrument antisubventions « distorsives », en améliorant le contrôle des investissements étrangers dans les actifs stratégiques ou en modifiant enfin son regard sur la concurrence internationale, notamment chinoise, l'Europe a montré ces dernières années qu'elle savait évoluer. Elle doit désormais dépasser un cap, pour ne pas passer à côté des nouveaux marchés des nouvelles technologies qui ne cessent d'éclore, pour ne pas être évincée par des concurrents déterminés et conquérants, pour ne pas être la variable d'ajustement

adapter rapidement aux transitions écologique et numérique, réduire nos dépendances stratégiques et, enfin, bénéficier de conditions de concurrence

d'abord mettre sur pied un plan d'urgence pour envoyer un signal très clair aux entreprises européennes et leur donner de la visibilité. Tel est bien l'objet du projet de plan industriel vert, qui sera présenté par la Commission aux chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen de demain et après-demain. Nous soutenons ce plan, parce que nous y trouvons beaucoup d'éléments nécessaires à nos yeux pour préserver et même accroître la compétitivité de l'industrie européenne.

constitue le dernier volet de cette stratégie. Elle implique la mobilisation d'instruments autonomes et de défense commerciale qui soient à la fois protecteurs, dissuasifs et, j'ajouterai, assertifs : finie la naïveté, nous allons être offensifs ! Je pense en particulier à la protection du marché intérieur contre les subventions massives et les pratiques commerciales déloyales des États-Unis ou de la Chine.

En revanche, il ne faut pas que l'Union européenne soit une variable d'ajustement ; nous continuerons donc de nous battre contre cela et contre ce plan américain. plan américain. Ce paquet ambitieux combinera des flexibilités raisonnables en matière d'aides d'État, une accélération ainsi qu'une simplification de la politique industrielle et des négociations avec les États-Unis. Vous pouvez compter sur nous pour faire avancer une politique industrielle européenne digne de ce nom. Nous en

prises pour son application, la commission des finances a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 17 voix pour, 1 voix contre -à la reconduction de M. Nicolas Dufourcq aux fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance. demande du groupe Les Républicains, de la proposition de résolution relative à la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens de 1915-1918 présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution, par Mme Valérie Boyer, M. Bruno Retailleau et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 227). Dans la discussion générale, la parole est à Mme Valérie Boyer, auteure de la proposition de résolution.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a près de huit années, je poussais les portes du Sénat ; j'étais alors présente non pas dans cet hémicycle, mais dans les tribunes. Je veux saluer les représentants de l'association des Assyro-Chaldéens en France, le président Marius Yaramis, François Pupponi, Georges Oclin, les élus Tony Fidan et Jean Samat, le professeur Efrem Yildiz, le président du Seyfo Center, Sabri Atman, et tous ceux qui n'ont pu être à leurs côtés dans nos tribunes, mais Permettez-moi de saluer, plus particulièrement, le professeur Joseph Yacoub et son épouse Claire. Vous êtes les enfants, les rescapés d'une entreprise de destruction massive, d'un génocide. génocide. Il y a plus de onze ans, le Sénat marquait l'histoire en votant le texte que j'avais présenté au Parlement sur la pénalisation du négationnisme du génocide de 1915. Il y a près de vingt-deux ans, malgré les pressions diplomatiques, le Parlement votait la reconnaissance du génocide arménien. Je n'imaginais pas, à cette époque, siéger dans cet hémicycle et devoir de nouveau parler d'un génocide. Je tiens à remercier le président Larcher d'avoir inscrit à l'ordre du jour cette proposition de résolution relative à la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens de 1915-1918. Je veux aussi remercier, plus particulièrement, Bruno Retailleau, qui s'est toujours mobilisé sur ce sujet, ainsi que le président Hervé Marseille, qui a accepté de s'engager à nos côtés. Aussi, en ce 8 février 2023, j'espère que nous saurons nous rassembler pour une cause universelle, qui nous transcende, celle de la justice et des droits humains. Même si l'histoire est un perpétuel recommencement, elle ne doit pas être un renoncement éternel. Pour la première fois en France, la question du génocide des Assyro-Chaldéens fait l'objet d'un débat public, suivi d'un vote. Nous ne le disons pas suffisamment, mais oui, le destin de l'Occident et l'avenir de l'Orient sont intimement liés. Le sort des chrétiens d'Orient et des autres minorités, notamment les Yézidis, peut être considéré comme un prélude à notre propre sort. Aujourd'hui encore, les chrétiens d'Orient sont en danger de mort et nous sommes les témoins de ce massacre annoncé, et même revendiqué. Souvenons-nous du 8 juin 2014 : Daech en Irak et au Levant prenait le contrôle de la ville de Mossoul, l'ancienne Ninive, capitale des empires assyriens, qui comptait autrefois plus de 30 000 chrétiens assyro-chaldéens. Ces barbares ont provoqué la fuite de près de 10 000 chrétiens de cette ville dans laquelle les maisons appartenant à la communauté assyro-chaldéenne ont été marquées de la lettre, en référence au terme « Nazaréen », qui désigne les chrétiens. Ces derniers ont été sommés de se convertir à l'islam, de payer la jizya ou de quitter la ville sans rien emporter avec eux sous peine d'être mis à mort. Cette cité s'est vidée en quelques jours de toute sa population chrétienne. Selon l'Évangile de Saint-Luc, « s'ils se taisent, les pierres crieront ». Mais il sera trop tard. Et demain, qui parlera l'araméen ? Qui parlera la langue du Christ ? Cent huit ans après 1915, l'histoire bégaie.

ils sont islamistes aujourd'hui, mais la méthode reste exactement la même. Ce génocide revêtait différentes formes et n'épargnait rien : il était physique, culturel et cultuel. Plus de la moitié de la communauté, estimée à environ 500 000 membres, fut martyrisée.

Je veux le redire, nous avons un rôle de protection envers les chrétiens d'Orient, qui est l'héritage d'une longue histoire remontant aux Capitulations signées par François Iavec le sultan Soliman le Magnifique en 1536. La mémoire et l'histoire contribuent à l'identité des peuples. L'oubli et la négation portent atteinte au respect de la dignité humaine. Ne laissons pas la France faillir à son devoir historique et moral de protection des minorités chrétiennes, pour ne pas faire rougir l'histoire ! Il y a un siècle, le génocide des Assyro-Chaldéens-Syriaques a été ignoré ; il continue d'être méconnu, comme le sort des chrétiens d'Orient aujourd'hui. Malheureusement, au travers de ce texte, nous parlons autant d'histoire que d'actualité. Pour les chrétiens d'Orient, l'histoire bégaie : ils font toujours face à une volonté de les éradiquer, de les éliminer, de les effacer.

ainsi, de manière abjecte, les survivants des génocides. Ces propos font peser une menace, celle de poursuivre cette extermination. Hier comme aujourd'hui, nous sommes face à une communauté désarmée, petite en nombre, mais majestueuse par sa culture. Hier comme aujourd'hui, nous sommes face à un peuple qui devient le bouc émissaire d'une radicalisation instrumentalisée par ceux qui veulent imposer par la force et la violence un régime qui n'a rien à voir ni à faire avec la religion, mais tout à voir avec la conquête du pouvoir et l'assouvissement des pires instincts humains.

Si, comme le dit le Président de la République, la France veut regarder l'histoire en face, elle ne doit oublier personne. Ce manque de reconnaissance est sans doute dû au fait que la nation assyrienne est souvent méconnue. D'ailleurs, l'Europe n'a jamais placé le sort des chrétiens d'Orient au premier rang de ses priorités- et c'est regrettable -parce que ceux-ci sont minoritaires, parce que nous dépendons de certains pays pour notre approvisionnement énergétique, parce que l'Europe a mauvaise conscience en raison de sa lourde responsabilité dans les conflits qui ravagent le Moyen-Orient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. nous avons appris de nos erreurs, nous avons payé le prix de nos fautes. Et parce que nous sommes à la fois les protecteurs historiques des chrétiens d'Orient, mais aussi le pays des droits de l'homme, ces génocides du XX siècle comme du XXI siècle ne doivent pas rencontrer la passivité de la communauté internationale,

Hélas, nous ne pouvons que déplorer la passivité de l'ONU en termes de protection de ces minorités, victimes de tortures et de purification ethnique. C'est pourquoi il est impératif que la plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale (CPI) par la Coordination des chrétiens d'Orient en danger aboutisse. Ban Ki-moon, alors secrétaire général de l'ONU, affirmait le 20 juillet 2015 que les actions intentées contre les chrétiens pouvaient être considérées comme un crime contre l'humanité. Mais il s'agit aussi d'un véritable génocide, comme je l'avais dénoncé à l'Assemblée nationale. Ces génocides sont aussi la matrice de notre civilisation et nous obligent à agir au nom de l'histoire et des engagements de la France. Comme l'explique Joseph Yacoub, « ce génocide physique et cette spoliation des terres et des biens étaient accompagnés d'atteintes graves à l'héritage culturel ». Malheureusement, ces exactions se poursuivent. Comme aujourd'hui les Arméniens de l'Artsakh, les Assyro-Chaldéens se sont vus déposséder d'une grande partie de leurs lieux de vie, de culture et de mémoire. En tout, plus de 400 églises et monastères ont été ruinés. Plus de 250 000 Assyro-Chaldéens-Syriaques, soit plus de la moitié de cette population, ont péri des mains des Turcs et des irréguliers kurdes utilisés à ces fins. Aussi, notre texte a plusieurs objectifs. Nous demandons notamment au Gouvernement de reconnaître officiellement que l'extermination de masse, la déportation et la suppression de l'héritage culturel de plus de 250 000 Assyro-Chaldéens par les autorités ottomanes entre 1915 et 1918 constituent un génocide. Nous l'invitons aussi à condamner publiquement ce génocide et à faire du 24 avril la date de commémoration annuelle du génocide arménien et du génocide assyro-chaldéen. Et à ceux qui parlent de « concurrence des victimes », je réponds « universalité des victimes » et « universalité de la cause Rappelons-nous cette phrase d'Élie Wiesel : « En niant l'existence d'un génocide, en l'oubliant, on assassine les victimes une seconde fois. » Avec cette proposition de résolution, nous donnons l'occasion à la France d'inspirer ses voisins européens et, plus largement, les démocraties occidentales.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l'ont rappelé les auteurs de la proposition de résolution, la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens s'inscrirait dans la suite de celle du génocide des Arméniens de 1915, portée par la loi du 29 janvier 2001.

Nous portons tous la même appréciation sur ces moments tragiques de l'histoire. Bien entendu, il faut condamner les massacres perpétrés, entre 1915 et 1918, contre la communauté assyro-chaldéenne-syriaque, un peuple réduit, du fait de sa faible population contemporaine, mais riche de sa culture, et immense par les gloires qu'il assume ou qu'il rappelle ; un peuple poussé à la marginalisation et contraint à l'immigration un peuple ayant presque entièrement péri, sans que l'Europe s'émût et sans que nul y prêtât intérêt, plongé dans l'oubli et dans l'indifférence générale ; un peuple sans État, que le climat favorable aux nationalités, il y a de cela un siècle, a oublié, abandonnant à leur sort ses quelques milliers de survivants. Après s'être engagé à apporter des garanties pour la protection des Assyro-Chaldéens et d'autres minorités ethniques ou religieuses à l'intérieur des régions d'un empire ottoman alors démantelé, Paris a finalement rendu caduc tout accord intervenu. Or, à l'heure du règne des États-nations, sans son propre État, un peuple n'a point de salut. L'idéologie nationale qui cimente les États récemment constitués privilégie souvent, à l'excès, l'appartenance au groupe ethnique majoritaire. Entre l'émiettement en micro-communautés et un ordre étatique négateur des particularismes minoritaires, la France doit jouer le rôle de porte-étendard des États démocratiques et de protecteur des minorités. Néanmoins, avant de porter notre réflexion vers toute forme de reconnaissance, il est important de rappeler la controverse entourant la qualification de génocide et le rôle du législateur dans sa quête de la juste vérité historique. Rappelons que reconnaître des faits inventoriés par des historiens n'est pas refaire l'histoire, et l'on se gardera bien d'avoir des positions à géométrie variable. Si les Assyro-Chaldéens n'ont jamais connu, semble-t-il, le bonheur des « peuples sans histoire », leur massacre répond indiscutablement,, à la qualification de crime contre l'humanité. peut ou non retenir la dénomination de génocide, je ne souhaite pas que, sans consensus, nos actes mémoriels incitent à une guerre des mémoires et à une concurrence des victimes. Il y a eu, et il y a encore, tellement de malheurs, d'atrocités, d'exactions, de guerres et de conflits qui ont jalonné et jalonnent encore notre histoire ... Il faut donc qu'il y ait non pas concurrence, mais universalité des victimes. Nos indignations ne doivent pas être sélectives. Or, s'il nous appartient de reconnaître le génocide arménien, et désormais le génocide assyro-chaldéen, sur quel fondement refuserions-nous de reconnaître celui des Tutsis au Rwanda ? Et la liste est si longue ; scrutez l'actualité Néanmoins, la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens, dont le massacre fut, je le rappelle, avéré en son temps par la Société des Nations (SDN), doit constituer un jalon majeur pour la justice et la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes, au Moyen-Orient comme partout ailleurs dans le monde. Cet acte mémoriel ne doit pas stigmatiser, culpabiliser, exclure ou diviser les populations actuelles en qualifiant de génocidaires les descendants des coupables de ces exactions. Au contraire, les faits établis de manière définitive doivent faire l'objet d'une acceptation unanime et servir de fondement à une réconciliation. Si les souffrances des Arméniens ont principalement attiré l'attention de la communauté internationale au siècle dernier, ce texte va dans le sens des récentes évolutions en la matière. En effet, ce sont consécutivement l'Association internationale des spécialistes du génocide (IAGS), l'Allemagne et le Saint-Siège qui ont consacré l'extermination concertée des Assyro-Chaldéens par l'Empire ottoman de 1915 à 1918 comme génocide.

Son adoption avait en effet provoqué de graves tensions diplomatiques entre la France et la Turquie. Or, si le contexte ne doit pas interférer sur ce qui est juste, je doute que le moment soit opportun pour raviver les tensions entre nos deux États, alors qu'Ankara, endeuillée, fait face aujourd'hui à la plus importante catastrophe de ces quatre-vingts dernières années, laquelle nécessite tout notre soutien. C'est pourquoi le groupe RDSE, fidèle à sa diversité et attaché à la liberté de vote, s'en remet à l'appréciation de chacun de ses membres.

la culture est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Quand on veut détruire un peuple, on cherche à effacer son empreinte culturelle, à détruire tout ce qui peut ressembler à une architecture- des églises, des monastères

qui n'avait cessé au cours des âges, de génération en génération, de jeter des passerelles culturelles, y compris religieuses, entre toutes les communautés. Et c'était souvent le seul trait

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après le séisme qui a frappé la frontière turco-syrienne, je tiens à faire part de notre soutien aux peuples kurde, syrien et turc et avoir une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Il y a plus d'un siècle, la Première Guerre mondiale a pris fin. Ce conflit a été d'une ampleur et d'une violence jusqu'alors inconnues, qu'il est aujourd'hui difficile de se représenter. Cette guerre, qui aurait dû être « la Der des Ders », a fait près de 20 millions de morts. En massacrant ses enfants, l'Europe s'est suicidée, selon le mot de Romain Rolland. Même s'il a cessé depuis plus de cent ans, ce conflit continue de produire des effets. Cette guerre a en effet marqué la fin du temps des empires, tant en Europe qu'en Asie Mineure et au Moyen-Orient. Elle a également décimé les populations des plus grandes puissances du monde. Comme trop souvent dans l'histoire, une tragédie en a entraîné d'autres. Alors que les regards étaient fixés sur les combats du théâtre européen, la Turquie ottomane, engagée dans le conflit aux côtés de l'Allemagne, a profité de la guerre pour régler ses comptes en 1915, elle a perpétré un génocide contre les populations arméniennes. Alors que ce génocide a été maintes fois décrit et documenté, Ankara refuse toujours de le reconnaître. L'ampleur des massacres, leur caractère ciblé et systématique, ainsi que la volonté d'effacer ce peuple, sont pourtant indiscutables. Les Arméniens n'ont pas été les seules victimes des massacres perpétrés par la Turquie ottomane en cette année 1915. Les Assyro-Chaldéens ont, eux aussi, subi des déplacements forcés et des exécutions en masse. Cette population comptait un demi-million de personnes à la fin du XIX siècle. La moitié d'entre elles a disparu dans les massacres. À ne pas reconnaître le passé, on se condamne à le revivre. Les auteurs de la présente proposition de résolution rappellent à juste titre que les chrétiens d'Orient ont figuré parmi les premières victimes de l'État islamique. Nous ne devons pas laisser dans l'ombre ces crimes contre l'humanité. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui invite le Gouvernement à reconnaître le génocide perpétré par la Turquie contre les Assyro-Chaldéens.

Le second objectif est un objectif de protection : reconnaître ces massacres comme le génocide qu'ils constituent mettrait en lumière des populations qui étaient encore récemment victimes de persécutions. Cette reconnaissance mettrait ainsi en lumière à la fois les Assyro-Chaldéens et la menace qui pèse sur eux. La communauté internationale serait dès lors plus attentive à leur sort. Alliés de la Turquie, toujours candidate à l'entrée dans l'Union européenne, nous attendons de ce pays qu'il agisse dans le respect des valeurs humanistes. Or, après avoir acquis des S-400 russes, Ankara n'a pas hésité à éliminer une frégate française, ne l'oublions pas. Elle use du chantage migratoire contre l'Europe et bloque l'adhésion des pays européens à l'Otan. La Turquie n'hésite pas non plus à recourir à la force contre ses minorités et celles de ses voisins. Nous avons vu son action contre les Kurdes de Syrie en Irak. Ces agissements graves sont particulièrement préoccupants. Loin de reconnaître son passé, Ankara semble vouloir continuer d'effacer ce qui la dérange, selon un comportement que plusieurs régimes autoritaires ont adopté à travers l'histoire, toujours avec des conséquences funestes. Dans ces conditions et au regard de la longue histoire qui nous lie aux chrétiens d'Orient, il nous semble que la France doit contribuer à empêcher de nouvelles atrocités. de résolution défend utilement tant la mémoire des victimes concernées que la survie de leurs descendants. Les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires voteront donc en faveur de l'adoption de cette proposition

monsieur le ministre, mes chers collègues, qu'il me soit permis avant d'évoquer cet épisode dramatique de l'histoire du Proche-Orient, d'avoir une pensée émue pour les dizaines de milliers de victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, pour leurs familles et leurs proches, pour celles et ceux qui sont encore coincés dans les décombres, celles et ceux qui tentent de les sauver et celles et ceux qui désespèrent de revoir l'être aimé. Notre collègue Boyer et le groupe Les Républicains nous proposent d'adopter une résolution relative à la reconnaissance du génocide assyro-chaldéen. Permettez-moi d'abord de relever, comme l'a fait notre collègue Temal récemment, que lorsque nous proposons à la majorité sénatoriale de réparer par le droit une faute commise par la République, à l'endroit notamment des soldats fusillés pour l'exemple de la Grande Guerre, le groupe Les Républicains nous accuse de vouloir réécrire l'histoire mais que la chose ne vous pose nullement problème quand il s'agit de proposer lois et résolutions mémorielles sur l'histoire d'autres pays. C'est différent ! C'est une contradiction de plus. Pour notre part, nous n'avons pas de problème de principe avec le vecteur législatif comme outil de politique mémorielle. L'histoire est une matière mouvante, une construction à la fois scientifique, sociale et politique, qui évolue avec le temps, à mesure des découvertes, de l'étude des archives et de l'évolution du point de vue que portent sur elle les sociétés. Avec toute la rigueur scientifique indispensable à l'exercice, il me paraît normal que le Parlement se penche sur notre histoire. La période sur laquelle vous nous invitez à réfléchir compte parmi les plus dramatiques et les plus douloureuses de notre histoire. Parmi toutes les horreurs de la Première Guerre mondiale, celles qui ont été commises par l'Empire ottoman, puis la Turquie naissante, continuent de hanter nos mémoires. Aux XIX et XX siècles, l'Empire ottoman regroupe une population majoritairement musulmane, ainsi qu'un ensemble de minorités chrétiennes de diverses églises schismatiques, considérées comme des citoyens de second ordre, notamment les Arméniens, les Assyriens, les Syriaques, les Yézidis, les Chaldéens ou les Grecs pontiques, fréquemment victimes d'exactions et de massacres. En 1909, le mouvement nationaliste des Jeunes-Turcs arrive à la tête de l'Empire et cherche à imposer sa politique de turquisation, qui prend de l'ampleur avec le début de la guerre mondiale. Pour éviter la fracturation de l'Empire et la révolte des populations chrétiennes, soutenues par l'ennemi russe, les autorités turques musulmanes ont mis en place un véritable plan d'extermination de ces dernières. Au total, entre 1 et 1,5 million de personnes est tué dans ces massacres et des centaines de milliers d'autres Ces abominables massacres, dont les racines sont à la fois politiques, identitaires et religieuses, ce qui est un peu trop oublié dans l'exposé des motifs de la présente proposition de résolution, sont communément reconnus sous l'appellation de « génocide arménien » et ont fait l'objet d'un consensus historique très large et d'une reconnaissance politique importante, qui n'incluent malheureusement toujours pas la Turquie. Si la réalité des populations non musulmanes et non turques de l'Empire ottoman dépasse la seule population arménienne et s'il ne fait pas de doute que toutes ces populations ont été massacrées sans distinction par le pouvoir ottoman, peut-on néanmoins distinguer et parler de « génocide assyro-chaldéen » suit la définition du génocide de la convention des Nations unies de 1948, il faudrait pour cela que les Assyro-Chaldéens représentent un même groupe national, ethnique, racial ou religieux. Pareille affirmation ne fait pas l'objet d'un consensus historique et mériterait un colloque bien plus savant que notre débat du jour. Les populations assyriennes, syriaques et chaldéennes, même si elles partagent une langue commune, peuvent-elles être considérées comme un même peuple ? Ce n'est pas le choix retenu par les très rares pays qui reconnaissent distinctement la logique génocidaire des massacres et qui, comme la Suède ou les Pays-Bas, distinguent les Assyriens, les Syriaques les Chaldéens, mais aussi les Grecs pontiques, également massacrés et étrangement absents du périmètre de la présente proposition de résolution. Vous l'aurez compris, faute d'un consensus historique plus large, il nous semble que la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 inclut dans son spectre l'ensemble des massacres perpétrés par l'Empire ottoman au cours de la période concernée et satisfait donc largement toutes les demandes de la présente proposition Mais si tel n'est pas l'avis de la majorité sénatoriale, pourquoi ne pas présenter une proposition de loi pour compléter ou préciser la loi de 2001 plutôt qu'une Ne niant pas le caractère systématique des massacres perpétrés contre les populations non turques, mais considérant que la réflexion qui sous-tend la présente proposition de résolution n'est pas encore aboutie, et n'oubliant pas un contexte géopolitique complexe et un contexte humanitaire dramatique en Turquie, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires

d'avoir une pensée émue pour la Turquie et la Syrie et pour toutes les familles des plus de 10 000 victimes, selon le dernier décompte, qui ont péri dans les terribles séismes survenus dans leurs pays.

dans les régions au sud-est de l'actuelle Turquie et au nord-ouest de l'Iran, a été déplacée de force et certains de ses membres tués par les forces ottomanes entre 1915 et 1918. Les estimations sur le nombre total de morts varient entre 180 000 et 275 000. La question arménienne a longtemps occupé le devant de la scène ; peu de chercheurs se lançaient à l'époque sur le sujet. assyro-chaldéen. de résolution à visée mémorielle n'est qu'un texte purement déclaratif qui, s'il était adopté, n'aurait qu'une portée symbolique ; ce n'est pas un véhicule législatif susceptible d'entraîner une quelconque amélioration pour les milliers de chrétiens encore persécutés en Orient ou pour les descendants des Assyro-chaldéens

: « Comme en 1915, les victimes sont chrétiennes et les bourreaux musulmans. » Mais c'est vrai ! Par une extension de sens, cela revient à sous-entendre que les musulmans sont toujours les coupables. Cet amalgame renforce tous les sentiments négatifs qui existent à l'égard de la religion musulmane. Il est dommage qu'un sujet historique d'une telle complexité soit passé au travers d'un filtre déformant et simplificateur. Pour l'opinion publique, l'enjeu est simple : reconnaître un fait. Pourtant, la réalité est plus complexe : précautions sémantiques sur la définition du génocide, agendas politiques, concurrence mémorielle, relations diplomatiques multilatérales ... Nous ne sommes pas face à un noeud gordien qu'il faudrait trancher avant de repartir examiner un autre texte, le coeur serein. La politique mémorielle passe aussi par des actions qui peuvent avoir un caractère symbolique très fort, telles que des discours de chefs d'État. Le Président de la République Emmanuel Macron a déclaré La France, c'est d'abord et avant tout ce pays qui sait regarder l'histoire en face, qui dénonça parmi les premiers la traque assassine du peuple arménien. En réalité, le problème est ailleurs. Le président de l'Union des Assyro-Chaldéens de France (UACF) le fait comprendre clairement : les Assyro-Chaldéens se sentent oubliés. C'est une question d'égalité dans la reconnaissance, au-delà de celle de la vérité Au cours des années 1990, avant les premières recherches universitaires sur le Sayfo, les groupes de la diaspora assyrienne ont commencé à communiquer auprès de différents gouvernements. En décembre 2007, l'Association internationale des chercheurs sur le génocide a adopté une résolution reconnaissant le génocide assyrien. Le parlement suédois en 2010, puis les parlements arménien et néerlandais en 2015 et le parlement allemand en 2016 ont suivi. Toutefois, très peu d'États se sont engagés dans cette voie. On ne peut donc pas dire que la majorité des États ait accepté cette démarche ni qu'elle fasse consensus, puisque Israël et le Royaume-Uni ont refusé de voter une disposition similaire à celle que nous examinons aujourd'hui. Néanmoins, nous sommes depuis longtemps les soutiens et les amis des chrétiens d'Orient.

Il faut le dire : la France s'est toujours montrée solidaire des minorités opprimées du Moyen-Orient, que ce soit par la voix des membres du clergé, comme l'abbé Eugène Griselle ou l'archevêque de Paris, ou par celle d'élus, à l'instar de Denys Cochin, député de Paris et membre de l'Académie française.

Plus récemment, devant des défenseurs des chrétiens d'Orient, le mardi 31 janvier dernier, à l'Élysée, le Président de la République a annoncé le doublement des fonds destinés à soutenir les écoles chrétiennes au Moyen-Orient. Créé en 1920, ce fonds avait déjà soutenu 174 l'année dernière. « Soutenir les chrétiens d'Orient est une mission historique » et un « engagement séculaire de la France » a dit le Président de la République. Nous considérons que ce texte, dont l'exposé des motifs comporte des raccourcis et des parallèles

permettez-moi de dire quelques mots sur le tremblement de terre qui a ces dernières heures frappé la Turquie et la Syrie. En effet, ce 6 février, ce sont bien deux séismes, à neuf heures d'intervalle, d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter pour le premier et de 7,5 pour le second, avec comme épicentre la ville de Gaziantep, qui ont durement frappé les populations. À l'heure où nous parlons, plus de 11 000 morts sont d'ores et déjà recensés. Le nombre de blessés sera beaucoup plus important, vous l'imaginez bien. bien. Une course contre la montre est engagée pour tenter de retrouver les survivants, pris au piège des débris et lourdement affectés par des températures glaciales. À jamais, ces femmes, ces hommes et ces enfants seront marqués et touchés dans leur chair et dans leur âme par ces événements. Je veux, au nom de mon groupe, leur dire tout notre soutien et leur adresser nos sincères condoléances. Nos pensées sont tournées vers eux. La France est aux côtés des peuples turc et syrien, qui souffrent. J'associe bien évidemment nos concitoyens qui, de par leur histoire familiale, vivent en France, leur pays, qui sont angoissés par la situation et attendent des nouvelles. Enfin, je souhaite souligner la formidable solidarité internationale, qui a su se mobiliser pour agir. La France y prend toute sa part. Nous ne pouvons que remercier le Président de la République et saluer Mes chers collègues, ce mercredi 8 février 2023 est un moment attendu, pour ne pas dire espéré, et ce depuis bien longtemps- trop longtemps -par la communauté assyro-chaldéenne.

Oui, en ce mercredi 8 février 2023, il nous revient par nos votes de reconnaître leur histoire, douloureusement marquée par ce génocide. En cet instant, je souhaite dire quelques mots à celles et ceux qui s'interrogent sur le sens même du vote de cette proposition Je pourrais leur répondre que l'histoire de France est aussi celle d'un pays qui a toujours pris ses responsabilités pour protéger les chrétiens d'Orient. Je ne vais pas ici revenir sur l'ensemble de cette histoire commune, car le temps me manquerait, mais il faut le rappeler. Je souhaite également saluer l'action des présidents de la République, MM. François Hollande et Emmanuel Macron, qui, ces dernières années, ont eu à agir en accueillant des réfugiés assyro-chaldéens menacés de mort par Daech. Ils ont été à la hauteur de leur mission : nous devons les en remercier. Je pourrais également leur dire que la France a toujours fait le choix de protéger les minorités, ainsi que leur culture et leur histoire, sans distinction religieuse, que ces peuples soient de confession chrétienne, musulmane ou juive. Je pourrais enfin ajouter que, il y a plus de deux siècles, la France a fait le choix de devenir la patrie des droits de l'homme et de faire de l'universalisme son champ de réflexion et d'action permanent. Je me dois aussi de leur dire que la position de mon groupe n'est pas de peser au travers de cette proposition de résolution sur les relations diplomatiques avec la Turquie, la Syrie ou tout autre État du Moyen-Orient. Notre position ne s'inscrit pas non plus dans une quelconque logique de guerre de civilisation ou de matrice civilisationnelle, car l'une comme l'autre sont infondées et mortifères. Mes chers collègues, il ne s'agit pas pour le Sénat d'écrire l'histoire. C'est le rôle et la mission des historiens : laissons-les travailler. Néanmoins, le rôle du Sénat est bien de prendre acte de l'histoire et ici l'histoire est claire le génocide assyro-chaldéen par la puissance ottomane est avéré. Près de la moitié des 500 000 Assyro-Chaldéens ont été pourchassés, tués, massacrés ou supprimés par la puissance ottomane.

Elle se transmet de génération en génération, comme j'ai pu le constater. Elle voyage au gré de l'exil, des villages montagneux à la nouvelle capitale des Assyro-Chaldéens qu'est devenue Sarcelles, dans mon département du Val-d'Oise. ans après les premières arrivées d'Assyro-Chaldéens dans notre pays, devenu aujourd'hui le leur, nous pouvons saluer leur amour de la patrie, leur volonté farouche de faire grandir la République sans jamais oublier leur histoire, leur culture, leur langue, ainsi que leurs frères et soeurs qui sont encore là-bas.

Pour conclure, permettez-moi de reprendre les mots de Victor Hugo, qui siégeait sur les travées du Sénat, celles-là même où vous êtes assis, chers collègues : « Servir la patrie est une moitié du devoir,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, Walter Benjamin disait que le progrès humain ne peut se réaliser tant que la justice n'est pas rendue aux victimes des persécutions. Nous devons aux morts du génocide arménien, à leurs souffrances et à leur mémoire qu'une instance juridique internationale établisse les faits et les culpabilités. Comme les Juifs de la Shoah, les Bosniaques de Srebrenica et les Tutsis du Rwanda, les victimes du génocide, des déportations et des spoliations perpétrés par l'Empire ottoman en 1915, qu'elles soient arméniennes, grecques pontiques ou assyro-chaldéennes, doivent être reconnues par un tribunal pénal international sous mandat de l'Organisation des Nations unies. La recherche historique a montré depuis longtemps que le génocide arménien de 1915 est non pas un accident, mais la phase paroxysmique d'une administration de plus en plus criminelle des minorités religieuses et ethniques par l'Empire ottoman. Pour bien en mesurer l'importance, il faut rappeler que les Arméniens, Grecs, Juifs, Syriaques, Assyriens et Chaldéens représentaient plus de 19 % de la population ottomane en 1914, contre 0,2 % aujourd'hui. La construction de l'État turc moderne s'est nourrie de la persécution des minorités religieuses et ethniques. Les minorités chrétiennes ont été éliminées les premières. Puis vint le tour de celles qui furent considérées comme incompatibles avec l'identité nationale fondée sur le sunnisme et la turcité. Ainsi, une violente campagne antisémite aboutit à l'expulsion des Juifs de Thrace en 1934. Progressivement, les minorités religieuses issues de l'islam subirent elles aussi la persécution : chiites, alaouites et alévis. N'oublions pas les massacres commis contre les communautés alévis de Sivas en juillet 1993 et de plusieurs quartiers d'Istanbul en mars 1995. Enfin, comment oublier le destin funeste du peuple kurde, auquel le traité de Sèvres promettait un territoire autonome au sein duquel seraient reconnus des droits pour la minorité assyro-chaldéenne ? Son article 62 prévoyait en effet que sa mise en oeuvre devait « comporter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou religieuses dans l'intérieur de ces régions ». On sait ce qu'il advint de ce traité, que la France et le Royaume-Uni s'empressèrent de remplacer par celui de Lausanne, signé en 1923, qui organisa leur tutelle sur les possessions ottomanes au Proche-Orient et abandonna l'Arménie et les Kurdes à leur triste sort. Pis, ce traité permit la réalisation de ce que la partie turque qualifia de « stabilisation de l'homogénéité ethno-religieuse » et qui se traduisit dans les faits par l'expulsion d'un million et demi de Grecs de Turquie. Un tiers d'entre d'entre eux moururent avant d'atteindre les côtes grecques. Ce génocide des Grecs de Turquie ne doit pas non plus être oublié. C'est vrai ! Le traité de Lausanne a posé les bases de l'identité religieuse et ethnique du nouvel État turc. Un ministre de la justice de Mustafa Kemal Atatürk déclarait en 1930 « que tous, les amis, les ennemis et les montagnes sachent bien que le maître de ce pays, c'est le Turc. Ceux qui ne sont pas de purs Turcs n'ont qu'un seul droit dans la patrie turque : c'est le droit d'être le serviteur, c'est le droit à l'esclavage ». La France accepta tout, jusqu'à l'opprobre de céder à la Turquie, en juin 1939, le sandjak d'Alexandrette qui appartenait au territoire de la Syrie placée sous son mandat. Les 50 000 Arméniens, Grecs et Assyriens qui y vivaient prirent eux aussi le chemin de l'exil. de résolution, chers collègues, vous écrivez que « la France [a un] devoir historique et moral de protection des minorités chrétiennes d'Orient ». L'histoire nous enseigne malheureusement qu'elle ne l'a assumé que lorsqu'il pouvait satisfaire ses ambitions géopolitiques. Ce pragmatisme sans scrupule a considérablement affaibli ces communautés et en tout premier lieu celle des Assyro-Chaldéens, sans doute parce que la diversité de ses composantes, linguistiques, religieuses et ethniques la rendait encore plus fragile. Minoritaires parmi les minorités, persécutés parmi les persécutés et oubliés parmi les oubliés, les Assyro-Chaldéens n'ont cessé de subir les conséquences des bouleversements de l'histoire tumultueuse du Proche-Orient. La France, en reconnaissant le génocide arménien, qui ne concerne pas seulement les Arméniens, ne les a pas ignorés. Le mérite de cette proposition de résolution est de les associer plus distinctement à l'hommage rendu à tous les morts du génocide. La parole est à M. François Bonneau.

de l'instruction publique, transcrit les témoignages non seulement des victimes des atrocités de l'Empire ottoman, mais également des témoins oculaires. Alors que le tribunal de la Conférence de la Paix allait se prononcer sur le sort de cet empire déchu, son objectif était de faire connaître aux juges et à l'opinion publique l'asservissement, depuis des siècles, de chrétiens en Arménie, en Asie Mineure et en Syrie. En apportant ces témoignages, Joseph Naayem a souhaité graver dans le marbre la mémoire d'un peuple oublié. Il dit notamment J'ai à coeur d'établir le martyrologe d'un petit peuple, le plus intéressant, mais en même temps le plus abandonné, issu d'un grand empire de la plus ancienne civilisation du monde, dont le pays fut, comme l'Arménie, le théâtre des abominations turques dont les hommes furent tragiquement assassinés, les femmes, les enfants et les vieillards déportés au désert, pillés, martyrisés, soumis aux pires outrages. Ce peuple, c'est le peuple assyro-chaldéen. Durant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman décimait les populations arméniennes et les Assyro-Chaldéens, se rendant coupable de crimes contre l'humanité. Alors que l'un a été reconnu comme un génocide par la loi du 19 janvier 2001,

Il est reconnu dans le cas d'« actes, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Il peut s'agir d'un meurtre, d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, d'une soumission intentionnelle ou encore d'un transfert forcé d'enfants. Exodes, famines, déportations, viols, enlèvements, acculturation ou encore conversions forcées, voilà ce qu'ont subi les victimes assyro-chaldéennes de 1915 à 1918. Les massacres se déroulaient dans un périmètre très vaste : en Anatolie orientale, en Perse et dans la province de Mossoul, c'est-à-dire dans des lieux identiques à ceux où périssaient les Arméniens. Dans les deux cas, les nationalistes turcs souhaitaient éliminer les groupes non turcs et non musulmans de zones géographiques trop sensibles en les exterminant, en les dispersant ou en les déportant, afin d'homogénéiser l'Empire. Nul doute n'est permis : il s'agit bien d'un génocide. Nous sommes la France, le pays des droits universels, des droits de l'homme et du citoyen. Il y va de notre héritage, il y va de notre honneur de reconnaître ce génocide, en dehors de toute autre considération vis-à-vis du pays qui nie ces faits. Reconnaître publiquement et officiellement est une manière de ne pas occulter ces drames et ces massacres perpétrés à l'encontre de ces grands oubliés dans l'ombre des victimes arméniennes. Alors que les yeux du monde étaient tournés sur les événements de la Première Guerre mondiale en Europe, l'Empire ottoman a assurément su profiter de la conjoncture pour se débarrasser de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui ne demandaient qu'à vivre sur ce sol, comme leurs ancêtres depuis des temps immémoriaux. Sous la Turquie de Mustapha Kemal, les communautés assyro-chaldéennes ont été marginalisées. Ces questions ne pouvaient émerger au niveau collectif ou sur le plan politique en raison du nationalisme ambiant, turc comme arabe. Ce n'est qu'à partir des années 1980 qu'un débat s'est ouvert sur ces massacres, par le biais des enfants et des petits-enfants de la diaspora. Les autorités turques actuelles, issues de l'ancien Empire ottoman, refusent d'admettre leurs responsabilités et leurs actions génocidaires face à des minorités culturelles et religieuses. S'il est toujours nié par Ankara, au même titre que le génocide arménien, le massacre des Assyro-Chaldéens est aujourd'hui reconnu par la Suède, par le Parlement néerlandais, par l'Australie, par l'Arménie ainsi que par le Vatican. En 2023, il n'est plus acceptable que l'État turc refuse de se confronter à cette cruelle réalité historique, celle qui a coûté la vie à plus de 250 000 Assyro-Chaldéens en trois ans et réduit en esclavage des milliers d'autres. L'heure est venue d'une reconnaissance officielle de ces crimes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un génocide. Cette reconnaissance est indispensable et pourra permettre de créer une lame de fond, afin qu'un jour le gouvernement turc l'admette à son tour.

L'hostilité à l'égard de ces populations reste prégnante dans ces régions. À titre d'exemple, l'engagement politique et militaire de la Turquie avec l'Azerbaïdjan contre les Arméniens au Haut-Karabakh a mis à nu le passé et a révélé la manière, particulièrement grave, Comment ne pas rapprocher le massacre des Assyro-Chaldéens du XX siècle des tueries meurtrières des chrétiens et des yézidis d'Irak et de Syrie par Daech ces dernières années ? Les motivations et le contexte politiques sont certes différents, mais les conséquences sont similaires : des événements laissant des milliers de morts et qui ont ébranlé les fondements mêmes de la vie de l'ensemble de ces communautés. Dans ces deux cas, des groupes minoritaires religieux ont été ciblés de manière systématique en raison de leur foi et ont été soumis à des violences extrêmes. Ils ont été condamnés sans autre issue que celle de fuir ou de mourir. La reconnaissance du massacre des Assyro-Chaldéens en tant que génocide et la condamnation des actes de Daech contre les populations chrétiennes et yézidies sont des premiers pas importants pour faire face à ces crimes contre l'humanité et pour prévenir leur répétition à l'avenir. Oui, cela fait plus d'un siècle, mais ne nous disons pas qu'il est trop tard, car ce serait une erreur, une nouvelle erreur. Il n'est jamais trop tard pour rendre hommage aux victimes. En reconnaissant l'existence du génocide, nous honorons leur mémoire et leur sacrifice, leur permettant ainsi de maintenir leur identité culturelle et religieuse. Il n'est jamais trop tard pour préserver l'histoire. En reconnaissant le génocide, nous nous assurons que ses leçons ne sont pas effacées et que les drames du passé ne finiront pas dans l'oubli. Il n'est jamais trop tard pour offrir une justice aux victimes. Reconnaître le génocide, c'est en quelque sorte apporter une forme de réparation pour la souffrance et les sacrifices du peuple assyro-chaldéen. En somme, il n'est jamais trop tard pour éveiller les consciences. La reconnaissance ne pourra que sensibiliser l'opinion publique aux causes et aux conséquences de ces tragédies et inciter d'autres pays à prendre des mesures en ce sens. La démarche engagée par Mme la sénatrice Valérie Boyer et M. le président Bruno Retailleau est importante. Il ne s'agit pas de procéder à une réécriture de l'histoire, mais de reconnaître, de mettre les mots sur la vague meurtrière qui s'est abattue sur ce peuple du Proche-Orient. Le groupe Union Centriste, dans sa très grande majorité, votera pour la proposition de résolution. Mes chers collègues, je ne peux que vous encourager à soutenir ce texte. Il ne s'agit pas d'un simple vote, mais d'un acte réparateur, d'un acte de justice pour se souvenir de ce génocide

à l'heure où les populations de Turquie et de Syrie pleurent les victimes du séisme du 6 février ou cherchent encore des survivants dans les décombres, je voudrais d'abord adresser les pensées et les condoléances du Gouvernement aux peuples de ces deux pays.

concerne le projet de résolution qui nous est présenté ce soir, je voudrais attirer l'attention de votre Haute Assemblée sur l'amalgame malheureusement réalisé entre les questions mémorielles de l'Empire ottoman, qui relèvent du travail des historiens, et la situation contemporaine des chrétiens d'Orient, en faveur de laquelle nous sommes bien évidemment pleinement engagés. Les questions mémorielles nécessitent un travail de recherche approfondie permettant d'éclairer des faits historiques. Elles ne peuvent être débattues qu'à la lumière d'une telle analyse, qui participe au travail de mémoire sur les événements tragiques de notre passé. Afin d'établir la reconnaissance du crime de génocide, une lecture juridique est en outre nécessaire. La définition du crime de génocide renvoie en effet à un corpus juridique international précis, désormais établi par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ainsi que par les statuts des tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda ou pour l'ex-Yougoslavie et, bien sûr, de la Cour pénale internationale. Nous devons aussi tenir compte des différences de contexte et nous ne pouvons examiner cette proposition de résolution sans tenir compte de l'exposé des motifs qui la justifie. En 1915, les victimes des massacres auxquels se réfère le projet de résolution étaient toutes chrétiennes. Il en va différemment des événements des dernières années. Si les chrétiens ont, à l'évidence, été la cible des atrocités de Daech, des membres d'autres communautés ont été visés, comme les yézidis, les chiites ou encore les sunnites que l'organisation terroriste considérait comme déviants. De fait, c'est parmi les musulmans que les victimes de Daech sont les plus nombreuses. Nous avons besoin, pour protéger les chrétiens et les membres des autres minorités, de l'engagement des gouvernements concernés, mais également des populations musulmanes majoritaires qui, elles aussi, souffrent du terrorisme. Affirmer ainsi qu'en 2023 les victimes sont chrétiennes et les bourreaux musulmans relève d'une vision partielle et partiale de l'histoire à laquelle le Gouvernement ne peut souscrire.

Ce soutien est pluriséculaire et s'inscrit dans une longue histoire d'amitié avec les communautés chrétiennes d'Orient. Celle-ci remonte à l'accord dit des Capitulations, conclu entre François I et Soliman le Magnifique, qui confia en 1536 à la France le privilège et la responsabilité de la protection des catholiques de l'Empire ottoman. Si ces instruments juridiques ne sont plus en vigueur, sauf en Israël et en Palestine, la France conserve une responsabilité politique et morale vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Comme l'a dit le Président de la République à plusieurs reprises, ce passé nous oblige. Voilà ! Notre pays continue donc d'agir en faveur des chrétiens d'Orient et des autres minorités du Proche et du Moyen-Orient. par fidélité à des populations qui sont proches de nous et par cohérence avec son engagement en faveur des droits de l'homme, en particulier de la liberté de religion. Il le fait également par conviction. Le maintien de la diversité religieuse au Moyen-Orient est une condition indispensable à son évolution vers la paix, la stabilité, la tolérance et la prospérité. C'est pourquoi notre pays s'engage pour toutes les minorités au Moyen-Orient. Ainsi, la France a pris l'initiative d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, en mars 2015, avant d'organiser, en septembre de la même année, une conférence internationale pour la protection des victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient. Le plan d'action issu de cette conférence reste une boussole pour la communauté internationale. De plus, la France agit aussi par elle-même. Je veux ici mentionner quelques exemples de notre action. Tout d'abord, nous apportons un appui financier important pour prévenir des violences religieuses dans la région.Entre 2015 et 2022, la France a ainsi mobilisé le fonds de soutien aux victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient, à hauteur de 39,4 millions d'euros, pour financer 123 projets, notamment en Irak et en Jordanie. Ces projets portent sur la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, le soutien psychologique, les moyens de subsistance et la stabilisation- déminage, relance économique, conservation du patrimoine culturel. À la demande du Président de la République, nous avons créé un fonds pour les écoles d'Orient. Revenons à 1915 ! Il présente la particularité d'être cogéré et cofinancé par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et l'OEuvre d'Orient, organisation non En 2022, ce fonds a distribué 4 millions d'euros d'aides aux écoles confessionnelles diffusant la francophonie au Proche-Orient, en particulier au Liban. Son action sera reconduite pour le même montant en 2023. La violence peut être aussi immatérielle. C'est pourquoi la France s'engage également dans la protection du patrimoine culturel et religieux des chrétiens d'Orient. Je pense au soutien que nous apportons à l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (Aliph). Il s'est trompé de fiche ! Cela a permis de mener une trentaine de projets de réhabilitation du patrimoine en faveur des chrétiens d'Orient À Mossoul, au coeur d'une ville meurtrie par des mois d'occupation par Daech, Aliph finance la restauration de l'église chaldéenne Al-Tahira, dont le dôme s'était effondré. La France s'engage aussi sur son territoire en faveur de la préservation du patrimoine culturel des chrétiens d'Orient. Il a par exemple été décidé, en 2022, de créer un nouveau département au musée du Louvre consacré aux arts de Byzance et des chrétientés orientales. Je voudrais aussi citer notre action de lutte contre l'impunité des crimes commis en Syrie et en Irak. Nous soutenons la documentation des crimes et violations des droits de l'homme commis par Daech et l'ensemble des belligérants et mettons tout en oeuvre pour que les responsables de ces crimes puissent être traduits devant des juges. Enfin, nous entretenons un dialogue au plus haut niveau politique avec les autorités religieuses. Ainsi, lors de l'audience papale du président de la République à l'occasion de sa visite au Saint-Siège, les 24 et 25 octobre 2022, il a notamment été question du maintien de la diversité religieuse et de la protection des chrétiens d'Orient. Le Président de la République, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et nos ambassadeurs sur le terrain rencontrent les chefs religieux chrétiens et musulmans et les encouragent

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.